l'ordre du jour appelle l'examen des crédits de la mission Relations avec les collectivités territoriales Arctique 45 45 bis 45 terre 45 quater 46 et du compte spécial avances aux collectivités périodes tutorial du projet de loi de finances pour 2023. La parole est à monsieur Charles Guené, rapporteur spécial de la commission des finances pour sept minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, je vais commencer par présenter les principales dispositions des articles rattachés à la mission qui concentreront l'essentiel de nos débats, l'article 45 propose diverses mesures, en lien avec la répartition de la DGF hein, en 2023 et des fonds de péréquation horizontale, les principales avancées sont les suivantes : en 1er lieu une hausse de 320 millions d'euros des composantes quoi triste la DGF, dont 200 millions d'euros au titre de la dotation de solidarité rurale un abondement complémentaire de la DGF, d'un montant équivalent a été prévu en première partie de façon à ce que cette année la progression des dotations de péréquation, ne soit pas financée par écrêtement des dotations forfaitaires, c'est une bonne chose, puisque cela marque un retour à l'esprit initial la péréquation verticale qui avait été quelque peu dévoyé ces dernières années l'article propose également une réforme de la DSR, avec le remplacement du critère de longueur de voiries utilisées dans le calcul des attributions versées au titre d'effraction péréquation et cible de cette dotation par un critère de superficie pondéré par un coefficient densité et un coefficient de population conformément aux délibération du CFL il prévoit également la neutralisation à nouveau en 2023, les effets de la réforme des modalités de calcul de l'effort fiscal prévu par la loi de finances pour 2022 nous avions suffisamment souligné l'an dernier le caractère inabouti de cette réforme, on ne peut donc qu'approuver cette mesure, mais la méthode qui consiste à adopter une réforme à l'aveugle pour ensuite en suspendre l'application 2 ans de suite laisse dubitatif en août 2 évolutions modalités de répartition du fonds de péréquation des ressources intercommunales le FPIC répondant à des recommandations que nous avions formulées dans notre rapport de contrôle qui ont consacré à à ce dispositif sur qu'ils il est prévu d'étendre sur 5 ans, le mécanisme de garantie de sortie en cas de perte d'éligibilité à un renversement afin de renforcer la visibilité des élus sur l'évolution de la ressource et de supprimer le critère d'insuffisance d'effort fiscal agrégé déterminant l'inéligibilité à un renversement. L'article 46 prévoit une augmentation de la dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité et pour la valorisation des aménité rural avec une majoration de 1 1000000 d'euros de l'infraction Natura 2000, une majoration de 200000 euros de l'infraction parcs nationaux et enfin une majoration de 4 millions et demi d'euros de la fraction parcs naturels régionaux. L'examen de l'article à l'Assemblée nationale a donné lieu à de nouveaux apports en 1er lieu les conditions des déchets milité seraient en infraction parcs nationaux, nos sondes assoupli puisque la dotation pourra désormais bénéficier aux communes dont le territoire est situé en tout ou partie dans un parc national et non plus aux seules communes dont le territoire terrestre est, en tout ou partie, y compris dans un coeur de parc national cette extension de la j'humidité concernerait environ 200 communes qui percevra alors une part forfaitaire de 3000 euros la 2ème modification vise à étendre l'éligibilité de la fraction parcs naturels régionaux à l'ensemble des communes dont le potentiel financier par habitant est inférieur au double du potentiel financier moyen par habitant des communes de la même strate et non plus des seuls communes dont des seuls communes dont le potentiel financier est inférieur à celui de la strate cette modification permettra ainsi d'assurer une harmonisation des critères financiers de Dish militer pour toutes les fractions de la notation. Par ailleurs, d'autres modifications sont intervenus pour modifier la répartition de la dotation pour titres sécurisés pour maintenir l'un des PEL comme une nouvelle ou encore pour que les préfets tiennent compte du caractère écologique des projets pour la fixation des taux de subventions accordées au titre de la DETR ou de la ces ces modifications vont dans le bon sens seulement cependant, il me semble important de rappeler le contexte économique actuel, l'inflation a atteint un niveau historique en 2000 22 et devrait se poursuivre en 2023, les collectivités territoriales ne sont pas épargnés par cette inflation qui a des répercussions tant sur leurs charges de fonctionnement que sur leurs dépenses d'investissement dans ce contexte un effet ciseau étant anticipé et pourrait générer un repli de l'auto-financement et de ce fait, de l'investissement des collectivités afin de soutenir les collectivités les plus en difficulté face à cette hausse de charge l'article 14 de la première loi de finances rectificative pour 2022 a prévu un nouveau prélèvement sur recettes visant à compenser partiellement au bloc communal Léo générés par la revalorisation du point d'indice, ainsi que la hausse des prix de l'énergie et de l'alimentation, ce dispositif ne concerne cependant que les collectivités du bloc communal et la hausse des charges, intervenue en 2022, or le contexte persistants d'inflation en 2023 continue de peser sur les finances des collectivités dont certaines font état d'une grande qui a inquiétude pardon pour finaliser leur budget primitif 2023 face à la hausse des dépenses énergétiques et envisage même la fermeture de service public un nouveau filet de sécurité a été intégrée au texte qui nous a qui nous a été transmis et que nos travaux ont permis de considérablement simplifié et renforcé en parallèle de ces dispositifs exceptionnels, les crédits de droit commun de la mission doivent permettre normalement de poursuivre le soutien à l'investissement des collectivités territoriales, je vous remercie pour votre attention. La parole est à monsieur Claude Raynal, à la fois président de la commission des finances et rapporteur spécial sur cette mission. Monsieur le président, madame la la ministre que je salue et félicite chers collègues dans le projet de loi de finances pour 2023 les autorisations d'engagement de la mission diminue de 636 millions d'euros à périmètre courant, tandis que les crédits de paiement progresse de 20 millions d'euros par rapport à elle a LFI 2022 cette diminution en autorisations et la conséquence d'un effet de périmètre, résultats de l'extinction de dispositifs ponctuels en 2022, notamment une baisse de 159 millions d'euros au titre la compensation des frais de gestion des régions et de celle du dispositif de compensation Ekoué des départements et de la non reconduction d'abondement exceptionnel 303 millions d'euros d'amende demain exceptionnelle en 2022 au titre là 250 millions d'euros au titre du plan Marseille et 20 millions d'euros afin d'améliorer l'attractivité de la Seine-Saint-Denis, retraité de ces mesures exceptionnelles les à eux de la mission connaissent une hausse de 108 millions d'euros qui s'explique essentiellement par la création de la dotation de compensation aux régions pour 91 virgule 3 millions d'euros, des frais de gestion de la CVAE commun à la suppression de la CVAE prévue par l'article 5 du PLF 2023 cependant, cette hausse à périmètre constant

à périmètre constant, c'est-à-dire retraitement fait des effets de périmètre susmentionnés les a eus enregistre donc une baisse de près de 176 millions d'euros et non une eau de 108 millions d'euros, et le S&P accuse une baisse de 140 millions d'euros et non une hausse de 20 millions d'euros, sans tenir compte de ces baisses intervenues en 2023 qui résulte en réalité de niveau exceptionnellement haut en 2022 les crédits des principales dotations sont stables depuis plusieurs années, ainsi la DETR est maintenu à 1 milliard la décide à 570 millions d'euros et la DPV à 150 millions d'euros, en revanche, la DTS enregistre une légère hausse, permettant de pérenniser le déploiement de nouvelles stations de recueil des Titres sécurisés qui a été rendue possible par l'abondement exceptionnel intervenue en première loi de finances rectificative pour 2022, d'un montant de 10 millions d'euros, la dotation biodiversité enregistre également une hausse puisqu'elle est portée à 30 millions d'euros, un AE et CP, soit 5,7 millions d'euros de plus qu'en 2022, cette nouvelle augmentation permet de porter à 4 euros l'attribution par habitant pour la appart naturel régional et de renforcer les autres fractions de la dotation le texte transmis par l'Assemblée Nationale prévoit une nouvelle hausse de 4,3 millions d'euros pour tenir compte, ne n'assouplissement des critères d'éligibilité à la fraction parc naturel régional cette baisse globale des crédits en tenant compte des effets de l'inflation va donc peser sur les investissements des collectivités qui sont par ailleurs confronté dans ce contexte inflationniste à une hausse de leurs charges de fonctionnement, ce double effet sur leurs ressources d'investissement et sur leurs charges pourrait ainsi générer une contraction de l'investissement local qu'il conviendra de surveiller durant l'année à venir enfin sur le programme 122 Concours spécifiques et administration, les crédits alloués à la reconstruction, à la suite de la tempête Alex diminue un eux mais augmente en CP afin de tenir compte des engagements antérieurs et et du rythme d'avancement des travaux, comme les années précédentes, et malgré ce constat de baisse des crédits en valeur, nous vous proposerons d'adopter les crédits de la mission, de même que ceux du compte de concours financiers avances aux collectivités territoriales, par ailleurs et à la suite du contrôle que nous avons mené cette année sur les dotations d'investissement, la commission a adopté 3 amendements qui seront débattues aujourd'hui, ils sont issus des constats que nous avons pu établir pendant nos travaux et des remontées qui nous ont été faites par les Hug locaux concernant surtout l'information relative à l'emploi de ces dotations d'investissement, le premier amendement et vise à instituer une obligation de consultation des présidents de conseils départementaux sur l'octroi de la dotation de soutien à l'investissement des départements, cette mesure serait de nature à institutionnaliser le dialogue avec les présidents de conseils départementaux en matière de décide, ça se fait dans beaucoup de départements tout de même et à favoriser la convergence des priorités nationales et locales quant au projet à soutenir le 2ème amendement a pour objectif de renforcer l'information des membres de la commission DETR sur l'emploi de la décide, au même titre que l'information actuellement mises en place pour la ce dispositif permettrait aux membres de la commission DETR d'avoir une vision exhaustive de l'emploi des subventions décident et décident dans leur département, le dernier amendement vise à renforcer l'information des membres de la commission DETR sur les demandes de subventions éligible mais finalement non retenue, permettant ainsi d'accroître l'information des élus sur les choix opérés par le préfet en matière d'attribution de subventions, cette mesure permettrait par ailleurs aux élus de mieux cerner les critères de sélection retenue par le préfet de vérifier évidemment le respect des priorités que la Commission a fixé d'éclairer son jugement sur les taux minimaux et maximaux de subventions à prévoir nos collectivités sont au coeur de l'investissement public et elles sont en première ligne pour aider nos concitoyens leur service publics doivent être préservés, a fortiori dans un contexte économique difficile, ils nous reviennent nous assurer qu'elles seront soutenus dans cette période et ce soutien peut et et doit prendre plusieurs formes : les aides exceptionnelles certes mais pas au détriment des dotations budgétaires annuelles et des concours financiers classiques, je vous remercie de votre attention. Merci monsieur le Président, rapporteur. La parole est à monsieur Loïc Hervé, rapporteur pour avis de la commission des lois pour 3 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le président de la commission des finances, mes chers collègues, comme en 2018 donc, fait rare, la commission des lois à cette année, et émis un avis défavorable à l'adoption des crédits de la mission Relations avec les collectivités territoriales, qui témoignent d'une grande inquiétude chez les élus locaux que les sénateurs de notre commission des lois ont très majoritairement souhaité exprimer en envoyant un message clair. Dans le contexte de défiance tout d'abord, si la première ministre a acté l'absence de sanction dans le nouveau dispositif de contractualisation financière l'insertion d'une telle disposition dans un texte adopté par la voix de la laine, il a 3 de l'article 49 de la Constitution, a créé un inutile climat de défiance que de temps et d'énergie perdus. Un contexte de perte de marge financière également, en raison d'une part de l'amoindrissement tendancielle des pouvoirs de décisions des collectivités en matière fiscale et d'autre part, de l'inflation qui ronge d'autant les capacités financières des collectivités territoriales, à cet égard la revalorisation annoncée de la DGF se traduira en réalité par une baisse en volume et les dispositifs de compensations financières en matière énergétique, ne semble pas avoir fait totalement leurs preuves dans ce contexte, la mission RCT que nous examinons aujourd'hui est-elle à la hauteur des craintes et des inquiétudes exprimées par les élus, notamment la semaine dernière à l'occasion du congrès des maires, la commission des des lois, a répondu par la négative, constatant que les crédits inscrits à l'échelle de la mission enregistre une baisse particulièrement regrettable de 12,84 % en autorisations d'engagement, le programme 119 qui concentre les crédits alloués au soutien à l'investissement des collectivités territoriales, connaît une diminution notion de 13,4 % en autorisations d'engagement du à l'extinction de plusieurs dispositifs, dont la non reconduction d'un abonnement de la décide à hauteur de 303 millions d'euros en 2022, ce retour au statu quo ante ne saurait nous satisfaire car il se traduira par une diminution en volume de 19,9 % de ses dotations dans ces conditions, inquiète du défaut de soutien de l'État à l'investissement local qui représentent une part déterminante du total de l'investissement public dans notre pays, la commission des lois a estimé que le fléchissement de la pluie, l'État aux collectivités territoriales, pourrait porter un coup fatal à nombre de leurs projets d'investissement au bénéfice de ces observations, notre commission des lois a donc émis un avis défavorable à l'adoption des crédits inscrits au titre de la mission, elle a malgré tout et heureusement et quand même adopté 5 amendements que j'aurais l'opportunité de vous présenter au moment de leur examen, je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur, la parole est à monsieur Guy Bénard Roche pour le groupe écologiste solidarité territoire pour cinq minutes. C'est le président. Merci, je confesse d'entrée de jeu comme en groupe ne pensent pas voter le budget de cette mission, sauf à constater des modifications significatives qui pourraient lui être apportés par les amendements or Loïc Hervé vient parler que nous soutiendrons et par ce que nous avons nous-mêmes déposé, bien sûr, il y a la stabilité apparente dans le contexte d'inflation mais surtout madame vie Dist, vous semblez avoir perdu de vue l'importance des éléments financiers et du levier financier majeur qu'il représente, non seulement dans la péréquation des moyens en local, mais aussi et surtout dans l'investissement local particulièrement en milieu rural avec les impératifs de la transition écologique, le projet de loi comporte de nombreuses missions qui s'attelle au soutien financier des collectivités territoriales et c'est au moins cela qui assure une certaine cohérence à ce projet de loi de finances et qu'il réduit le moyen des collectivités et de leur autonomie fiscale corollaire de leur libre administration. Ou compensation qu'elle serait en droit d'espérer c'est récurrent dans toutes les missions que vous avez porté, je ne suis pas le seul à regretter ce que mon collègue Loïc Hervé, qualifie de mouvement tendance. Ciel de réduction des marges de manoeuvre fiscale des collectivités territoriales et de leurs groupements, il a eu l'occasion de rappeler que la Cour des comptes, elle même, a estimé que la décomposition des ratios d'autonomie financière montre qu'il repose désormais davantage sur la fiscalité nationale que sur la fiscalité locale propre. Après les tergiversations parlementaire sur la CVAE l'arme du 49 3 avenir que vous utiliserez une nouvelle fois empêche totalement une visibilité essentiel pour les acteurs locaux, j'ai déjà pu aborder l'importance que nous devrions. Des on Mathias d'une gouvernance plus sereine au développement d'une démocratie plus forte localement et cela doit s'accompagner de moyens notre groupe porte une réelle vision de la gouvernance locale qui s'oppose à celle du gouvernement, en particulier sur le poids de l'autonomie fiscale mais aussi de leur gouvernance, nous avons de nombreuses reprises critiqué entre autres la mainmise du préfet sur les collectivités et nous continuera de le faire, ce pouvoir discrétionnaire dans l'attribution de Ford, soutien à ce pouvoir sur de nombreuses agences locales sanitaire ou environnemental, depuis la loi 3DS tout ceci lois n'bien trop de civils. Sur principal de contrôle de légalité et le rapproche d'un administrateur local il reste comme toujours dommageable que les collectivités restent à la porte de financement, alors même que l'avènement de la haine c'était. Avait été annoncé comme gage d'efficacité. Gage de guichet unique accompagnant les collectivités cette lotion de guichet unique fait écho aux mais France service que l'État a voulu mettre en place pour répondre aux attentes légitimes de nos concitoyens, particulièrement ceux qui se retrouvent les plus démunis face à une numérisation massive et rapide des services publics, mouvement qui je le rappelle, encore une fois, n'a rien de sacrificateur en tout cas pour les 13 millions de nos concitoyens, souffrant d'électro-le financement de ces maisons, la question du partage de la charge liée à la dématérialisation des services publics restent trop floues. D'un point de vue, plus précis, nous accueillons favorablement un amendement plus importante de la dot assure biodiversité, même si nous exprimant des réserves quant au bout d'alité d'attribution il filer des mentors la priorisation des concours financiers de l'État à la transformation écologique et urgence et toute action concrète dans cette voie est un pas de plus vers une réelle transition écologique, même si l'éco-conditionnalité Saab rester à tabou nous impressions, le niveau des aides aux communes forestières, victime de scolytes, mais là encore, même si ces subventions sont nécessaires, elle reste le reflet de l'absence de prévention dans les politiques publiques de ce gouvernement, la diminution du nombre de personnes de l'ONF, alors que les dangers sur les forêts sont de plus en plus prégnant et plus qu'un mauvais signal. C'est de la mauvaise gestion, Madame la Ministre, nous sommes satisfaits de voir la dotation politique de la ville stabiliser afin de répondre aux besoins des communes les plus en difficulté, au sortir de la crise sanitaire. Beaucoup de projets locaux en attente doivent pouvoir reprendre, nous regrettons cependant l'inadaptation évident de la dotation forfaitaire pour la délivrance des titres de sécurité mais dans ses missions, comme dans le reste du PLF, l'État ne prend pas assez la mesure de l'importance et de l'imminence des besoins des collectivités territoriales, acteurs primordiaux de la transition écologique comme pour la question des transports Doria dans ce texte. Le permet d'envisager des battements, renforcement des mobilités du quotidien. m'étonner l'intervention présidentielle de dimanche soir, sur le besoin de RER dans les métropoles après l'absence de soutien du gouvernement jeudi par exemple, pour avancer sur les amendements liés au versement mobilité, sénateur des Bouches-du-Rhône, j'en profite également pour dire que j'aurais sincèrement sur ma fait sur le volet transport alors que le projet le peu logements sur le plan Marseille en grand, lui, hé bien, fait bien partie de ce PLF pour terminer, je dirais que la dissonance habituel entre les déclarations et les moyens problématique qu'elle crée et nourrit le sentiment de défiance du local envers le National que la période du quoi qu'il en coûte 100 bien loin et que les difficultés locales sauf de nouveau échappé à ce gouvernement, les demandes étayées, des associations d'élus des institutions locales sont pourtant bien là en tout cas pour dans le groupe, le, le compte n'y est pas, c'est pourquoi nous nous associera certains abonnements et que nous présente des améliorations qui, faute d'être tu ne nous permettront pas de voter ce budget. Merci, cher collègue, la parole est à monsieur Didier Rambaud pour le groupe RDPI pour six minutes.

Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le président de la commission des finances, mes chers collègues, nous débutons donc ce matin l'examen des crédits de la mission Relations avec les collectivités territoriales, cette mission est l'occasion de rappeler le soutien de l'État aux collectivités, mais aussi aux élus locaux, à l'heure où la guerre fait rage à l'Est de l'Europe, et où il doit faire face à une crise énergétique inédite, en effet, cette mission s'inscrit dans la continuité des actions que le gouvernement mène depuis 2017 avec une méthode claire celle du dialogue renforcé, comme l'a rappelé la première ministre au dernier congrès des maires de France, l'État doit être accompagnateur au service des projets des collectivités et des élus au plus près des réalités du terrain et des besoins de nos concitoyens au fondement même de nos politiques publiques dans son ensemble pour 2023, les crédits de cette mission s'élève à 4 20 28 milliards d'euros en autorisations d'engagement et 4 37 milliards d'euros en crédits de paiement, la baisse d'autorisations d'engagement que nous observons est liée à l'extinction de dispositifs ponctuel financés en 2022, à l'instar de la hausse exceptionnelle de des îles de 303 millions d'euros et du plan, Marseille en grand de 250 millions cette mission se compose de 2 programmes budgétaires ayant vocation à soutenir l'effort financier de l'État en faveur des collectivités territoriales, les 2 programmes de la mission poursuivent plusieurs objectifs : tout d'abord le maintien du niveau des investissements locaux dans le souci de protéger les marges de manoeuvre des collectivités en effet les dotations d'investissement traditionnel du programme 119 qui comprennent la des îles classique, la DETR, la DPV s'élève à près de 2 milliards d'euros en à eux et à 1,78 milliards d'euros en crédits de paiement après avoir été l'aiguillon de la relance économique dans les territoires conséquemment à la crise sanitaire puis économique, notamment à travers la, la, des exceptionnel, ces dotations d'investissement contribue également aux mesures rendues nécessaires par le changement climatique, le 2ème objectif de cette mission et l'accélération de la transition écologique tout en surmontant la crise énergétique actuelle le PLF pour 2023 prévoit d'augmenter d'un tiers les moyens consacrés à la dotation biodiversité qui avait, qui avait d'ailleurs été doublés en 2022, pour un montant de 30 millions d'euros les communes concernées ont un parc naturel régional ou une zone Natura 2000, la progression de la dotation pour la biodiversité vient en complément de la création d'un fonds Vert, d'un montant inédit de près de 2 milliards d'euros, ce fonds sera coordonnée de manière déconcentré sous la responsabilité des préfets, ce fonds financera ainsi 3 types d'action, le renforcement de la performance environnementale dans les territoires, le radar adaptation au changement climatique, l'amélioration du cadre de vie, concrètement, grâce aux fonds vers les collectivités bénéficieront d'aides pour la rénovation énergétique des bâtiments publics locaux, la gestion et l'extension des aires naturelles protégées, la création ou le développement des zones à faibles émissions le recyclage des friches la renaturation en ville, le tri et la valorisation des déchets, la prévention des risques inondations, effondrements glaciaire cyclonique incendies de forêt, recul du trait de côte et pour surmonter la crise énergétique, le gouvernement a annoncé un ensemble de mesures pour accompagner les entreprises, les associations et les collectivités territoriales de mécanismes, à savoir le bouclier tarifaire et l'amortisseur électrique électricité seront déployés dès le 1er janvier 2023 et concerneront directement les collectivités et leurs établissements, il représente un soutien financier, estimé à 2,5 milliards d'euros, témoigner de la solidarité envers les collectivités qui font face à des aléas climatiques, c'est aussi l'objectif du programme 122 Concours spécifiques et administration, il connaît une forte hausse de 25,5 pour 100 en lien avec l'abondement de la dotation de solidarité aux collectivités victimes d'événements climatiques ou géologiques et du fonds de reconstruction pour les Alpes-Maritimes de près de 50 millions d'euros, enfin, et l'un des derniers objectifs poursuivis par la mission et le renforcement de la santé financière des collectivités je salue d'ailleurs la hausse de la DGF de 320 millions proposés, financé par l'État et non par écrêtement des autres communes, elle viendra abonder la DSU et la DSR, cette, cette augmentation inédite depuis 13 ans permettra le maintien ou l'augmentation des dotations pour 95 % des communes avec l'objectif impératif de maîtrise de notre dépense publique, cette augmentation est un véritable geste à l'endroit des collectivités et des élus locaux, en définitive, les crédits de la mission permettront aux collectivités locales de conserver en 2023, une bonne visibilité sur leurs finances et sur leur capacité d'investissement dans un contexte économique particulièrement défavorable, par ailleurs, concernant le compte spécial avances aux collectivités territoriales les crédits demandés pour 2023 s'élève à 124 milliards d'euros, soit une hausse de plus 8 66 % par rapport à 2022 avant conclure, permettez-moi de saluer quelques mesures introduites dans les articles rattachés le renforcement très Net de l'effort pour les communes d'outre-mer qui aura augmenté de 42 % depuis 2019 les évolutions liées aux modalités de répartition du FPIC qui répondent aux Ores au combat des recommandations formulées par notre commission des finances, la prise en compte du caractère écologique des projets pour la fixation des taux de subvention fixée au titre de la DETR de la disent-ils, par les préfets ou encore le maintien de la dotation particulière, élu local là des pelles pour les communes nouvelles créées à compter du 1er janvier 2023, mes chers collègues, la mission RCT le compte financier avances aux collectivités territoriales et les articles rattachés se caractérise par la continuité de l'action de l'État pour accompagner toutes les collectivités locales dans les situations d'urgence et dans leurs investissements de long terme, il témoigne également de la sincérité de ce PLF au service des collectivités et des élus locaux en responsabilité autant que sous réserve des discussions ont été un moment mon groupe bien évidemment votera les crédits de cette mission. Merci, cher collègue. à la suite de la discussion, à part l'État Didier Marie pour le groupe socialiste, écologiste républicains pour 9 minutes.

Monsieur le président, madame la ministre, messieurs les rapporteurs, comme chaque année, nous examinons en seconde partie du projet de loi de finances, les crédits de la mission Relations avec les collectivités territoriales. Nous le faisons cette année dans un contexte particulier, celui d'un environnement économique et sociale particulièrement anxiogène, conséquence de la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine. Les maires que nous côtoyons sont inquiets, beaucoup voient leurs Budgets déséquilibrés difficile à boucler, avec l'explosion des dépenses d'énergie, le renchérissement des produits alimentaires, celui des marchés de travaux. Tous voient la précarité gagner du terrain et les centres communaux d'action sociale, multiplie les aides aux plus démunis. Il est regrettable dans ce contexte que le gouvernement est considéré les collectivités territoriales comme une variable d'ajustement de son budget plutôt qu'un élément moteur de résilience. Le gouvernement se targue de travailler main dans la main avec les associations d'élus, le dialogue serait permanent, fructueux, le budget co-construit mais alors Madame la Ministre, pourquoi toutes ces associations, s'alarme-t-elle les projets du gouvernement, tout simplement parce que celui-ci confond concertations et consultations dialogues et monologues horizontalité et verticalité. Ce n'est pas faute d'alerter le gouvernement, nous l'avons fait encore lors des débats budgétaires de cette session. Or, lors de l'examen du projet de loi de programmation des finances publiques, vous avez décidé d'une nouvelle génération, des contrats de Cahors, non seulement vous continuez de ne pas faire confiance aux collectivités. Mais vous les infantiliser en les menaçant de sanctions, en les privant de dotation d'investissement si elles ne réduisent pas leurs dépenses de fonctionnement. L'Assemblée nationale et le Sénat, vous ont dit non. Stop à ce climat de défiance. Mais vous insistez en réintroduisant ce dispositif à l'article 40 quater de cette seconde partie du projet de loi de finances, ceci est doublement inacceptable pour les collectivités, suspecté de dépenser à tort et à travers, alors que leur budget ne peuvent être en déficit et pour le Parlement que vous tentez de bâillonner, Madame la Ministre, nous supprimerons ce de nouveau ce carcan dans lequel vous voulez placer les collectivités. 2ème sujet : la CVAE après la suppression de la taxe d'habitation dont la compensation continue de poser problème, vous poursuivez votre stratégie de nationalisation des impôts locaux et de réduction des marges de manoeuvre des collectivités. C'est tout de même extraordinaire qu'à chaque fois que le gouvernement souhaite faire des cadeaux fiscaux, il ne le fasse pas avec ses propres impôts. Mais avec les impôts locaux, nous mettant ainsi sous tutelle ce faisant vous couper le lien entre les territoires et les entreprises. Quel maire, à l'heure de la sobriété foncière arbitrera en faveur d'une activité industrielle, source de nuisances potentielles sans retour fiscal face à un projet immobilier re-tributaire, ce n'est pas le vague Font national de l'attractivité économique des territoires dont les critères de répartition ne sont pas définies qui leur assurera. Vous nous assurer la main sur le coeur que son remplacement par une fraction de la TVA sera profitable à nos communes et départements mais ce qui sera profitable aux entreprises les plus importantes en 1er ne le saura pas pour les ménages, sur lesquelles vous allez faire peser l'impôt un impôt particulièrement pénalisant pour les familles modestes qui en paient proportionnellement plus que les plus aisés, un impôt volatile qui a certes progressé plus vite ces dernières années que la CVAE mais dont la tendance peut se retourner en période de stagnation ou de crise. Une majorité s'est exprimé au Sénat pour maintenir la CVAE. Ne faites pas fi de nos arguments ne passait pas, une fois de plus en force avec le Ne restait pas accroché à votre dogme du moins d'impôts et renoncer à votre politique de désarmement fiscal qui se fait au détriment des services publics et du plus grand nombre. 3ème sujet : l'inflation et l'explosion des coûts de l'énergie, nous le répétons, les conséquences de la guerre en Ukraine sur le coût de l'énergie pénalise lourdement de nombreuses collectivités et mettent en cause leur capacité d'investissement. Nombre d'entre elles ont déjà reporté des réalisations prévu et annoncé il y a 2 ans, lors des élections locales. Toutes font preuve de responsabilité et d'imagination pour réduire leurs dépenses courantes. Mais comment accepter de réduire l'éclairage public, au risque de l'insécurité, d'augmenter les tarifs de restauration scolaire de baisser les températures dans les écoles et les crèches. Le gouvernement annonce la mise en place d'un filet de sécurité, à l'origine, il devait concerner 22000 communes puis 12000 aujourd'hui 7000 au mieux. Le Sénat vous propose de l'élargir et d'en resserrer les mailles, nous aurions souhaité aller plus loin que le rapporteur général mais nous prenons sa proposition, reste à savoir si le gouvernement fera de même à cela s'ajoute l'inflation sur les produits alimentaires, les travaux d'entretien courants les fournitures diverses et l'augmentation du point d'indice, c'est la raison pour laquelle, Madame la Ministre, nous vous invitons à écouter le Sénat et à ne pas revenir sur le vote concernant la revalorisation de la dotation globale de fonctionnement pour l'indexer sur l'inflation. Vous proposiez 320 millions d'euros hors inflation, nous aurions applaudi mais cette augmentation d'1,47 % hé bien loin des 4 à 7 % d'inflation estimée par la Banque de France. J'en viens aux crédits de la mission proprement dite, divisé en deux programme 119 et 122 ils représentent environ 4 % du total des transferts financiers de l'État aux collectivités et connaissent une baisse de 12,84 % des crédits d'engagement baisse particulièrement regrettable au regard du contexte que je viens d'évoquer. Si la baisse des crédits du programme 122 s'explique en grande partie par la baisse des crédits alloués aux collectivités victimes d'aléas climatiques, ceux du programme sont 19 vont peser sur l'investissement local. Ainsi les crédits, les dotations de compensation vont une fois de plus baissé de près de 8 % en volume, confirmant l'érosion progressive des compensations des compétences passer. Les crédits de soutien à l'investissement local connaissent eux une baisse en valeur de 13,2 % et de 19,9 % en volume, certes, le gouvernement nous dira que ces baisses sont liés à l'extinction, dispositif exceptionnel mais était-ce bien le moment de réduire ainsi le soutien à l'investissement local. Pour ce qui concerne les articles rattachés j'attire votre attention madame la Ministre, sur les craintes de pertes de la DPE elle des communes nouvelles qui pourrait en freiner la création, nous déposerons d'ailleurs un amendement pour soutenir cette démarche et relancer le processus d'encouragement au regroupement. Enfin, nous reviendrons, comme chaque année avec le rapporteur pour avis de la commission des lois. Sur les modalités de décision de répartition de la décide, et de la DETR ainsi que du Fonds Vert pour en améliorer la lisibilité et l'association des élus, Madame la Ministre, nous arrivons aux limites du pouvoir d'agir des collectivités territoriales, leurs moyens leurs moyens d'action se dégrade, alors que les élus ont répondu à chaque appel à la rescousse du gouvernement lors des différentes crises que nous avons traversé depuis 5 ans, gilets jaunes Covid crise économique et maintenant la guerre, vous sortez le bâton plutôt que la carotte et vous décourager les élus. Le président de la République annonce un nouveau chapitre de la décentralisation, nous lui rappelons que décentraliser c'est lâcher du lest et non tenir en laisse les collectivités locales ont besoin de visibilité, de moyens de confiance en les régents tant en les bridant on alimente la grogne sociale, l'incivisme et on fragilise la démocratie. Madame la Ministre pour toutes ces raisons, et pour l'ensemble de son oeuvre envers les collectivités territoriales, nous ne voterons pas les propositions du gouvernement pour les crédits de cette mission, je vous remercie. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, 40 ans, c'est le bel anniversaire que nous aurions dû fêter cette année, celui de l'acte I de la décentralisation en 1982 ce sont une série de lois qui marque alors une rupture avec la tradition centralisatrice qui a constitué pendant des siècles une forte spécificité de l'organisation politique et administrative de notre pays de Charlemagne, Louis XIV à la Révolution française, jusqu', Napoléon notre histoire centralisatrice plus que jacobine a marqué la construction politique multiséculaire de notre pays, à l'inverse, 1982 acte de la volonté d'une administration décentralisée, déconcentrée de notre pays, posant comme principe que le renforcement de la liberté locale tout en maintenant les pouvoirs régaliens de l'État renforce l'incarnation des principes républicains, cette année, aurait donc dû être une année de joyeux anniversaire des libertés locales, elle restera comme leur marche funèbre ce nouveau budget rogne largement sur les finances des collectivités, votre gouvernement, Madame la Ministre, par un nouveau 49 3 à l'Assemblée nationale a pris l'option de faire fi des discussions, des parlementaires sur le sort de nos collectivités territoriales, la loi de programmation budgétaire 2023 2027 rejeté par l'Assemblée nationale durci ici au Sénat, trace une feuille de route austéritaire et ce projet de loi de finances en découle, concrètement, c'est bien une perte de 2 9 milliards d'euros pour les collectivités territoriales qui a été votée, soit 13 milliards d'euros de DGF retirer aux collectivités territoriales, depuis 2014 la colère des élus montent, Madame la Ministre, depuis quelques semaines, comme d'autres ici je suis destinataire de motion adoptée par les conseils municipaux de mon département concernant les finances locales et j'ai une pensée ce matin pour les communes de Pouille et les faire Saint Paul Violet Saint-Nizier-sous-Charlieu Lentini Saint-Germain Laval out Chatel ou encore Saint-André d'Daxon et tant d'autres, madame la Ministre, nos collectivités doit faire face à une situation sans précédent, avec une inflation à son plus haut niveau depuis 1985 le constat est là, les dépenses annuelles de fonctionnement ont et vont exploser de plus de 10 milliards d'euros en cascade, ce sont les capacités d'investissement des collectivités qui sont amputés par effet domino, c'est notre activité économique, nos richesses territoriale nos employes locaux qui sont menacés chez les artisans, les TPE-PME de nos départements et pour reprendre l'expression de notre collègue Fabien Genêt oui il va y avoir de la casse, si rien n'est fait ainsi, après 4 ans de baisse des dotations de 2014 à 2017, la réduction des moyens s'est poursuivie depuis 2017 avec le gel de la DGF et la baisse chaque année des attributions individuelles pour plus de la moitié des collectivités du bloc communal, Madame la Ministre, l'heure n'est pas, à savoir la faute à quelqu'un qui en a, nous en sommes là la réalité s'impose à nous, parlementaires, avoue, gouvernement et surtout aux dizaines de milliers d'élus locaux qui, au quotidien, ont l'impérieuse nécessité de devoir répondre aux enjeux de leur population de développement des services publics locaux de gestion de leurs collectivités face à un assèchement des moyens financiers de leur capacité à agir pour assurer leur mission d'amortisseurs de crise ainsi dans le cadre de l'examen de ce projet de loi de finances, vous avez souhaité la suppression de la CVAE à laquelle le Sénat s'est opposé vous proposer de nouveaux contrats de Cahors, qui s'applique à plus de collectivité, que la première génération, mais nous en reparlerons lundi prochain, depuis 2014 la baisse cumulée des dotations, je l'ai dit, a conduit à l'effondrement des investissements alors que les comptes de l'État n'ont fait apparaître aucune réduction de déficit à contrario du budget que vous nous proposez, nous proposons un budget viable pour nos collectivités qui font vivre la démocratie, nous saluons donc l'indexation par le Sénat de la DGF sur l'inflation, même si nous regrettons que cette mesure ne soit acté que pour l'année 2023, nous saluons la possibilité du remboursement du FCTVA sur l'agencement et l'aménagement de terrains, alors que le filet de sécurité 2022 décrié sur tous les bancs de notre hémicycle et, de fait, Morné nous actons la proposition sénatoriale pour 2023, même si nous pensons qu'il lui fallu une meilleure visibilité du dispositif plus compréhensible par l'ensemble des élus nous demeurons convaincus qu'il faut aller plus loin et j'aurai l'occasion avec les membres de mon groupe de pouvoir et revenir dans le débat sur nos amendements dans le cadre de cette mission, en somme, nous défendrons un véritable projet de libre administration pour les collectivités territoriales, convaincue qu'avec ou sans 49 3 les mesures votées ici seront retenus, je vous remercie. Merci, cher collègue. Dans la suite de la discussion, la parole est à Nathalie Goulet pour le groupe Union centriste pour 3 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, monsieur le président de la commission des finances, mes chers collègues, nous consacrons à ce budget, 8 heures de débats, Madame la Ministre, c'est plus que les affaires étrangères, la défense et l'aide au développement cumulés, vous voyez l'intérêt que porte le Sénat à cette mission, donc j'ai quelques minutes pour vous dire le désarroi des territoires ruraux comme le département de l'Orne, avec la gestion des dotations mais je ne suis pas la seule en faisant des déjà parlé ce matin, je pense que la DETR a beaucoup perdu de son caractère rural Madame la ministre et qu'à la fois, on est en pleine schizophrénie parce qu'à la fois on a besoin de de rendre éligible, un certain nombre de charges à la DETR et en même temps ces charges qui correspondent en réalité à des normes supplémentaires ne devraient pas être imputés à la DETR pour laisser cette cette dotation pour pour les territoires, je pense notamment aux airs des gens du voyage ou à la défense incendie qui sont des normes supplémentaires extrêmement lourde dans l'intérêt général et cetera qui finalement pèse sur la DETR qui, de ce point de vue-là perd évidemment de sa de sa disponibilité pour pour d'autres projets cette c'est un sujet qui me semble extrêmement important, d'autant que cette DETR et notamment le refus DETR n'est jamais très claire, et que il y aura des amendements pour demander que le refus de DETR comme de d'ici le soit soit alors on me dit : oh non, on l'a déjà voté plusieurs fois dans cette maison, on me dit que la motivation va créer des recours pour une fois qu'on dit que ça crée pas des charges nouvelles, c'est quand même une bonne nouvelle, donc on examinera ce type d'amendement, plus 100000 euros pour la commission DETR ça laisse beaucoup de dossiers échapper au contrôle de la commission commission en question et je consacrerai la minute qu'il me reste pour vous dire que, par ailleurs, la gestion du fonds Vert qui ne dépend pas directement de vous mais qui finalement correspond à une dotation supplémentaire ne devrait pas échapper non plus au au contrôle de la commission DETR ou devraient être distribués dans les mêmes conditions, parce qu'il y aura probablement des départements où les fonds disponibles seront au moins égaux ou supérieurs au montant des dotations, donc ça va créer évidemment un un appel : il n'y a absolument aucune raison que la distribution et que le que le la distribution de cette dotation échappent à ce contrôle, donc il y aura aussi dans les articles rattachés un certain nombre d'amendements sur ce sujet, donc évidemment c'est la mission Écologie mais en même temps ça concerne ça Keiser ne les les collectivités et donc, d'autant que ce fonds Vert, c'est un peu les galeries Lafayette et la Samaritaine parce que depuis quelques jours dans cette maison, chaque fois qu'on évoque une dépense on dit mais ce sera le fond Vert, ce sera le fond Vert et cetera, donc je pense qu'il va falloir, il va falloir quand même cerner tout ça, il me reste quelques secondes pour vous dire que Belhout en Houlme la chapelle aux moines Le Chatelier, la gaufrier, la lande Patry Land Isaac masser, est mort sur huit n'ont pas reçu encore les dotations du au filet de sécurité, je vois que j'ai le plein soutien du président de la commission des finances qui qui sait très bien que cette tribune sert à nos territoires merci madame la mise. Dans la suite de la discussion, la parole est à monsieur Stéphane Ravier pour le groupe des non inscrits pour 3 minutes. Monsieur Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, nous voilà arrivés à la mission la plus importante de notre projet de loi de finances, celle des relations avec les collectivités territoriales, je dis la plus importante, parce qu'en France 70 % de l'investissement public et porté par ces collectivités, malheureusement, ces dernières n'ont plus de marge de manoeuvre pour assurer ses investissements dans le contexte que nous connaissons la responsabilité en revient pleinement à ce gouvernement qui a creusé, plus de 600 milliards d'euros de dettes supplémentaires tout en obligeant les communes à l'austérité budgétaire avec la suppression de 11 milliards d'euros de leurs recettes issues de la taxe d'habitation et en proposant maintenant la suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de la CVAE vous espérez que les communes résolve à leur frais, le paradoxe du en même temps entre le quoi qu'il en coûte dispendieux issus des restrictions de liberté, de la période Covid la casse d'EDF et notre soumission à l'austérité budgétaire imposée par l'Union européenne à nos administrations publiques dans mon département, Madame la Ministre, les centres des villes et villages perdent leur commerce la pérennité des services publics encore existants et menacé les déserts médicaux progressent et les inégalités territoriales s'accroissent le gouvernement est incapable d'alléger la pression fiscale de l'État sur les entreprises françaises et les ménages mêlés aux fonctionnaires de Bercy trouve toujours en impôt local a supprimé les communes après l'hôpital sont la variable d'ajustement de votre politique budgétaire avec la loi 3DS les élus locaux ont compris que vous n'aviez pas d'ambition réformer ni à simplifier le mille-feuilles administratif et le mille-pattes fiscal vous misez tout sur les les pôles métropolitains sans réelle vision pour la ruralité pour laquelle vous annoncez des millions, certes, mais des millions de migrants, alors que l'objectif de 0 artificialisation nette crée des tensions vous rompez le lien d'intéressement entre industrie et territoires par la suppression de la CVAE les communes ne pourront pas participer à la réindustrialisation du pays, je reste convaincu qu'une partie de notre salut ne peut venir que d'une sobriété, voire d'une cure de désintoxication fiscale je vous soutiendrai pour la suppression des impôts locaux, quand on vous supprimerez des impôts d'État depuis 30 ans, les ressources des communes sont en baisse, et ça continue dans ce PLF les dotations de soutien à l'investissement local diminue de 20 % en volume dans un contexte inflationniste à cela vous ajoutez un nouveau critère écologique flou pour l'attribution des dotations d'équipement des territoires ruraux et dotation de soutien à l'investissement local, ce qui renforce l'illisibilité pour les élus locaux, je finirai en rappelant que les communes ne représente que 4 % de la dette publique, toutes les collectivités confondues 9 % seulement de plus, l'État a le droit d'emprunter pour financer ses dépenses de fonctionnement pas les communes, elles ont donc pas de leçon de jeu de gestion à recevoir, c'est bien à l'État obèse et gloutons de faire l'effort de réduire son train de vie, la proximité communal, c'est l'avenir, c'est efficace, démocratique, économique patriotique écologique en l'état, je ne voterai pas cette cette mission de budget 2023. Dans la suite de la discussion, la parole est à monsieur Jean-Pierre Corbisez pour le groupe RDSE pour cinq minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, je ne déposerai pas ma liste de courses pour mon département du Pas-de-Calais mon bassin minier natal mais j'accepterais de laisser quelques subsides à ma collègue Maryse Carrère qui luttent contre le loup et l'ours, mes chers collègues, les élus locaux que nous avons la charge de représenter, ont toujours su faire preuve de réactivité, de responsabilité et ont répondu présents pour accompagner l'État dans la crise sanitaire qui a frappé notre pays, j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, il est grand temps que l'État restaure la relation de confiance qui doit entretenir avec les collectivités territoriales et là ce n'est pas le budget que nous examinons aujourd'hui qui en sera la meilleure traduction au delà des effets de périmètre exposés dans le rapport de nos collègues rapporteurs, force est de constater que les autorisations d'engagement et les crédits de paiement stagne, voire baisse alors que nous collectivités doivent faire face un contexte inflationniste particulièrement difficile ah a bien peu encourageant quand dans le même temps, les mesures prises par le gouvernement contraint davantage chaque jour les marges de manoeuvre ou de nos territoires ainsi et quand bien même l'État compenserait à l'euro près les recettes fiscales issues de la taxe d'habitation, la CVAE il n'empêche que si leur autonomie qu'on réduit progressivement le levier fiscal, nous le savons tous est l'un des rares outils que peuvent actionner les élus pour se donner des marges de manoeuvre, notamment s'ils souhaitent pouvoir investir pour maintenir le dynamisme de leur territoire et aux compagnies son développement, mais aujourd'hui ils ne le peuvent plus dans l'ensemble, nous observons des velléités de contraindre les dépenses de fonctionnement des collectivités, c'est un véritable coup de poignard dans le dos, tandis que dans le même temps, les déficits de l'État s'envole, c'est un métissage d'infantilisation adressé aux exécutifs locaux, Madame la Ministre a rien de mépris, oserais-je dire, bien éloignée du lyrisme de d'un discours présidentiel appelant à une véritable décentralisation chiche, serait-on tenté de lui répondre, quand bien même pour le bloc communal, on constate une stabilité de l'enveloppe je donc pour doit malgré tout ça, c'est de susciter la croissance inédite de l'inflation cette année qui se poursuivra en 2023 se traduira par une contraction des Budgets locaux et donc à une moindre incapacité à investir, à à quand la décoration de la DGF sur l'inflation, réclamée par les associations d'élus. Petit motif de satisfaction malgré tout avec la revalorisation du budget consacré à la préservation de la biodiversité et son ouverture plus large aux communes situées dans le périmètre d'un parc national, le scrutin dont par ailleurs les amendements proposés par nos collègues rapporteurs concernant les procédures d'octroi des doutes ont d'investissement de l'État, dès lors qu'il renforce l'information des élus locaux sur les décisions prises par le préfet. Un point sensible car le recours aux appels à projets pour l'attribution d'un certain nombres de subventions, cause de réelles difficultés aux plus petites collectivités peu outillés pour y répondre, or il est de la responsabilité de l'État, de garantir l'égalité de traitement, soit en simplifiant les procédures soit en accompagnant mieux les communes dans la dans la constitution des dossiers quant à la compensation de la participation des communes aux missions de l'État, elle doit être renforcée dans une véritable logique de partenariat de coopération et non avec un esprit de contrainte ou de prescription, je pense bien sûr à l'épineuse question de la délivrance des titres de sécurité ou celle de la contribution des communes aux frais d'installation et de fonctionnement des agences France service, une initiative qui dans son esprit est louable, mais dont les modalités de mise en oeuvre, ont constitué pour moi un véritable affront aux communes. Chacune d'entre elles offrent un lieu d'accueil bien identifié par nos concitoyens et plutôt que de lancer un nouvel appel à projets, il aurait été plus simple, plus efficace et plus respectueux d'attribuer une dotation supplémentaire aux communes pour leur permettent de remplir ses missions les retours que nous avons des élus locaux au quotidien au contact de leurs habitants semble dire que France service n'est pas une réussite partout je cache que nos communes aurait su mieux faire, avant de conclure : terre aurait la demande formulée par le passe par le passé par mon groupe RDSE de pouvoir débattent d'un véritable projet de loi de finances dédié aux collectivités territoriales, sortie du PLF annuel comme le sont les dépenses de Sécurité sociale avec le PLFSS c'est à ce prix que nous pourrons enfin construire une relation équilibrée entre l'État et les collectivités et reprendre sereinement nos discussions sur la préparation d'un nouvel acte de décentralisation, les membres de mon groupe RDSE se pose Jojo n'auront donc en fonction de l'évolution des amendements de déposés ou adopté, je vous remercie. Merci, cher collègue. Dans la suite de la discussion, la parole est à monsieur Stéphane Sautarel pour le groupe Les Républicains pour cinq minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, en préambule, je veux vous saluer vous féliciter, Madame la Ministre, tout en notant que vous êtes la 5ème interlocutrice des collectivités territoriales en 9 mois, la mission Relations avec les collectivités territoriales, n'est qu'un volet des moyens provenant essentiellement de prélèvement sur recettes qui sont alloués aux collectivités, puisqu'elle vient compléter les 105 milliards de transferts financiers de l'État et les mesures d'un vrai filet de sécurité, telle que proposée par le Sénat, si elle ne comporte que 4,37 milliards d'euros, elle n'en est pas moins importante, malgré une lecture en trompe-l oeil au regard des évolutions de périmètre tout d'abord, je me réjouis de la création de la dotation de compensation aux régions des frais de gestion de la CVAE à hauteur d'un peu plus de 4 heures 11 millions d'euros en conséquence de sa suppression prévue à l'article 5, même si cette question méritera d'être débattue, le programme 119 enregistre de son côté une baisse substantielle les crédits de la à la déciles qui revient à son niveau de 2021, à savoir 570 millions d'euros, nous reparlerons du Fonds Vert vendredi qui interroge tant il semble ouvert les autres crédits DETR DPV DTS sont stables ou en faible augmentation sur la DETR, plusieurs amendements visant à mieux communiquer à mieux partager et à davantage associer les élus locaux et les parlementaires aux décisions seront proposées : je ne peux qu'y souscrire mais pour en revenir au crédit, on ne saurait se sa petite sphère de l'apparente stabilité des crédits de la mission alors que nous sommes dans un contexte inflationniste, ce qui va avoir pour conséquence une réduction de la capacité d'investissement des collectivités, au-delà des difficultés rencontrées à l'échelle micro par chaque commune, chaque collectivité la contraction de leurs ressources, notamment du fait de la désindexation si elle elle devait être confirmée, contrairement à nos votes des dotations générera au plan macroéconomique un effet récessionniste qui nous guettent déjà à bien des égards, l'hypothèse de croissance pour 2023 retenu par le gouvernement et de un ce chiffre faible et déjà optimiste déjà ramené par le FMI à 07 soit revu à la baisse si les collectivités territoriales qui ne représente en France que 19 % du total de la dépense publique, contre une moyenne européenne proche de 40 40 % mais assume plus de 70 % du total de l'investissement public se voient privés de leur capacité d'autofinancement en raison de femmes de ce fameux effet ciseaux qui fait se croiser la dynamique des charges qu'elles subissent et l'atonie de leurs ressources, car là, et bien le véritable sujet, celui de l'auto-financement des collectivités je ne cesse de le dire, par-delà les crédits de la mission cette situation me semble préoccupante et devoir faire l'objet d'un suivi, enfin, au cours de l'exercice 2023 et d'une clause de revoyure générale et effective au titre des articles rattachés 45 et 46, je me réjouis de l'accroissement de l'enveloppe des composantes quoi triste de la DGF et en particulier des 200 millions d'euros de DSR complémentaire, en revanche, je m'interroge sur l'évolution des critères de calcul la charge majeur des petites communes rurales concernent la voirie communale est essentielle pour toutes les mobilités s'affranchir de ce critère pour retenir celui de la superficie ne me semble pas répondre aux objectifs de la DSR que nous envisagions, à terme, de mieux prendre en compte la réalité du territoire car nombre de charges sont indépendantes de la population et sont liées au territoire, bien sûr, mais en l'espèce, cela ne semble pas juste et, surtout, dans cette hypothèse, ce n'est pas la superficie mais le potentiel financier superficiel qu'il conviendrait de prendre en compte, enfin, l'article 46 prévoit une augmentation de la dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité pour la valorisation des aménité rural la valorisation introduite de 5,7 millions d'euros, élargissement des communes éligibles sont appréciables mais encore limitée des amendements seront présentés pour aller plus loin, surtout, j'insiste sur la nécessité de prendre mieux en compte cette considération positive pour nos territoires qu'il conviendrait, non seulement de mieux valoriser dans cette mission, mais aussi au au-delà pour finir, il est évident que cette mission ne peut s'inscrire que dans un climat de confiance qui nécessite la suppression de l'article 40 Potter dont la réintroduction par le gouvernement ne peut être ni comprise ni admise au moment d'aborder une nouvelle étape de la décentralisation que nous appelons de nos voeux, avec une vraie confiance accordée aux territoires dans leur totale autonomie et la liberté d'administration je vous remercie de votre attention. là. Parole est à monsieur Dany Wattebled pour le le groupe les indépendants pour cinq minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Je souhaite tout d'abord salué le formidable travail du locaux leur noble mission les m'en première ligne face aux difficultés énergétiques et financières que nous connaissons leur dévouement envers leurs administrés Guy leur action au quotidien, même quand les moyens et les solutions viennent à manquer. L'État doit être à la hauteur de leur engagement et leur donner les moyens d'agir. Pourtant, la mission Relations avec les politiques territoriales voit ses crédits diminuer de 636 millions d'euros en le Kurdistan d'engagement, alors tu vois s'explique tout d'abord par la longue relation des dispositifs ponctuelles ou de centaines de mesures de soutien qui n'avait pas vocation à perdurer, il faut rappeler que l'année 2022 avec lundi exceptionnelle en termes de dotations par exemple le PLF 2 22 avait permis d'abonder la mission de crédit inédit, à l'image du plan Marseille en grand un projet d'ampleur qui avait mobilisé de 200 de 154 millions d'euros.

fait l'objet d'environ 4 milliards d'euros prévus en l'autorisation d'engagement soit c'est une baisse de 40 millions d'euros par rapport à l'an dernier. Le crédit destiné de soutien à l'investissement local sont certes bien moins important que lors du 22 mai elles reviennent à un niveau général des dotations observée entre 2018 et 2021 la quasi toute durée des crédits engagés dans le cadre du plan de relance ont été consommées notamment en matière de de Cécile des ciels rénovation thermique, j'en suis heureux, cela prouve que les élus ont su saisir les moyens supplémentaires proposés. Dans le programme qui réunit les crédits destinés aux concours spécifiques administration 4 milliards d'euros sont budgétés, soit une hausse de sortants, millions d'euros en cris de paiement qui s'explique notamment par les disques de soutien de l'État après la tempête Alex et les conséquences des inondations. Je l'ai dit, les crédits de la mission sont globalement stables et si donc on part aux années précédentes. Pourtant la baisse qu'ils connaissent par rapport à la année du 2022 ne peut nous satisfaire car toutes nos collectés vont connaître une réelle diminution de leurs ressources, puisque ces crédits ne font pas adossé au niveau de l'inflation et on sait que cette inflation en train de partir, c'est pourquoi, dans le cas de l'examen de la mission Relations avec les collectivités nous gros de retour, la baisse des crédits budgétés dans une période qui appelle au contraire à une intensification des dispositifs en leur faveur. Cette contraction de crédit envoie un mauvais signal aux élus locaux qui sont inquiets et qui nous sollicitent en ce sens, c'est la capacité à assurer le service public de proximité qui risque d'être menacée. Les collectivités jouent un rôle crucial en matière de développement économique de leurs territoires, rappelons-le, 70 % des investissements publics sont directement porté par le par l'échelon local, on parle là d'entreprise de professionnels d'artisans dont le rôle en matière d'emploi est crucial emploi local, en l'état actuel, le projet de loi de finances pour du le vingt-trois devait conduire à une diminution de quatre à six d'investissement des collectivités, je sais que nous en sommes tous fortement préoccupés et que nous serons vigilants dans les prochains mois sur les effets concrets des annonces gouvernementales en faveur de ces collectivités heureusement plusieurs dispositifs exceptionnels ont été mises en place récemment pour accompagner les collectivités, je pense notamment au filet de sécurité destiné aux communes et aux EPCI qui avait été voté dans le cas de la loi de finances rectificative pour 2022,

ce projet de loi de finances 2023 apporte des fonds pour les soutenir, nous allons étudier plusieurs amendements dont l'objectif de parfaire et d'euros c'est ce soutien à quand l'adossement de la DGS sur l'inflation souviens notamment l'amendement de bon sens porté par plusieurs collègues de nos mon groupe, les indépendants, son objectif de corriger les effets de seuil dont peuvent être victimes, certaines communes nouvelles dans le cas de l'attribution de la dotation de se hâter rural pour ces raisons, et malgré des réserves, le groupe, les indépendants, accueille favorablement ces crédits, relation avec les tutorial tout en appelant à poursuivre les dispositifs de soutien en faveur de l'échelon local face aux difficultés financières que connaissent nos élus. Merci, cher collègue, la parole est à madame Françoise Gatel pour le groupe Union centriste pour cinq minutes. Madame la ministre, monsieur le président, monsieur le rapporteur, alors bienvenue dans la chambre des territoires, voilà, je pense que ce soir vous repartirez tout à fait armés, Madame la Ministre, au-delà des des chiffres qui, qui sont l'objet de notre journée, parlons du fond, celui de l'inquiétude d'un monde qui vient chez les élus locaux qui doivent toutefois aux côtés de l'État, conduire le pays à bon port, ces élus sont au coeur de la ville de nos concitoyens face au doute, parfois à la colère, mais dans tous les cas, tenus de faire face et d'assumer des services qu'ils rendent, pour le compte de l'État et qui sont des services essentiels, car ils sont ceux de la solidarité, de l'égalité, madame la je suis sûr que vous partagerez mon propos les collectivités ne sont pas des caisses de charité, elles ne sont pas un problème, elles sont des solutions pour l'avenir de notre pays, la crise sanitaire la montrer donc quand elle demande c'est exigence pour assumer leur mission alors que vous dire aujourd'hui, alors je vais saluer les mesures de soutien de l'État aux collectivités, on ne peut pas découragé de bons gestes donc je salue tout cela toutefois, Madame la Ministre, nul ne saurait éluder la frustration des propositions si peu des disruptif du gouvernement, parfois trop complexe et pas à la hauteur, financières, car quand le contexte et si disruptive à cause d'une extrême fragilité des Budgets, notamment du bloc local et l'impossibilité d'amortir les 11 milliards du hausse de coût de l'énergie, on a un vrai sujet, car la crise énergétique va entraîner une autre crise énergétique avec le renoncement annoncé de 46 % des communes à mettre en oeuvre leur projet de transition énergétique mais aussi leurs projets d'investissement, or, Madame la Ministre, l'investissement des collectivités, c'est le moteur de l'économie et de l'emploi et si le moteur s'enraye l'économie tout sera fort, donc les crédits de soutien aux collectivités sont des dépenses d'investissement pour l'État, mais Madame la Ministre, pour les élus gémir n'est pas de mise, car les élus sont condamnés à réussir le présent et inventer l'avenir, c'est ce qu'ont fait plus de 2500 communes françaises qui, librement, se sont regroupés pour créer 787 communes nouvelles pour muscler pérenniser l'indispensable proximité toutefois le régime de dotation n'a cessé d'être chahuté depuis 2015 pour devenir par des vices cachés, c'est ainsi contre-alors Madame la je ne doute pas que la récente célébration à Château-Gontier, en Mayenne, où l'air est certainement très inspirant de l'initiative et de la responsabilité par le président de la République, je ne doute pas que cette inspiration vous inspirera alors Madame la Ministre, ma question est : claire choisiront nous dans ce monde mutants d'encourager soit de décourager pardon et de pénaliser sévèrement des élus courageux et lucide, qui ose entreprendre leur avenir ou choisirez-vous Madame la Ministre de plomber tristement leur avenir, faut-il rappeler qu'en 2014 80 communes de France n'ont pas eu de candidat aux municipales en 2020, elles étaient 110, l'heure est grave, Madame la Ministre, il ne faut pas se payer de mots, et ce n'est pas un hasard si, aujourd'hui, dans la chambre des territoires plusieurs groupes politiques que je salue, ont déposé un amendement pour soutenir cette révolution silencieuse que sont les communautés de communes et qu'il convient, Madame la Ministre, de ne pas décourager, je vous remercie. Merci, cher collègue. Dans la suite de la discussion, la parole est à Madame Sylvia Noël pour le groupe Les Républicains pour cinq minutes. Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, des de la transition écologique défis du numérique défis économiques et sociales démocratique sanitaire civique sécuritaire nos élus n'ont jamais été confronté à autant d'attente et de bouleversement en tout genre dans un contexte très mouvant et incertain ou leur pouvoir d'agir est entravée par une perte de pouvoir financier qui s'accroît d'année en année le vote des Budgets des collectivités territoriales pour 2023 ne fera pas exception, bien au contraire et s'inscrit dans un contexte inflationniste exceptionnel les collectivités sortiront de l'exercice 2022 avec une dégradation nette de leurs comptes surcharge résultant de la hausse du point d'indice, hausse des coûts énergétiques mais aussi alimentaires et des fournitures technique, ce qui réduira fortement leur épargne brute et contraindra leur capacité d'investissement, les conséquences de cette crise sont graves et menace directement le maintien d'une offre de services de proximité sur l'énergie, les élus locaux attendent une compensation des mauvais choix de l'État dont ils pâtissent, ils ne font pas l'aumône, ils attendent simplement du gouvernement la protection qui est dû à leur territoire et à leurs habitants, et on ne peut qu'espérer que le bouclier tarifaire proposée par le Sénat soit sauvegardés à l'issue de l'examen de ce texte, tant le dispositif proposé initialement par le gouvernement s'apparenter à une usine à gaz dont bien peu de collectivités auraient pu, au final, prétendre à ce contexte s'est ajoutée une augmentation de la masse salariale induit par la hausse du point d'indice de 3 et demi % qui ajoute une charge supplémentaire de 2,3 milliards d'euros pour nos collectivités, en dépit des efforts réalisés par les élus locaux pour tenter de contenir les dépenses et boucler leur budget en cette période de crise, l'exécutif leur a adressé un coup extrêmement brutale en réintégrant par la voix du 49 3 les contrats de Cahors, le message du gouvernement est clair, qu'importe, les associations d'élus locaux, l'avis du Sénat où le vote négatif de la majorité des députés, il imposera sa trajectoire de rigueur budgétaire aux collectivités et le mécanisme punitif aveugle qui l'accompagne ce dispositif qui concerne davantage de communes que la première édition, contraint les dépenses locales pour les 5 années à venir et s'apparente à une énième tentative de recentralisation, alors même que nos collectivités représentent 19 % au total de la dépense publique, contre 30 à 40 % en Europe, elles ont moins de pouvoir qu'ailleurs, alors qu'elles représentent 75 % des investissements tout l'enjeu est là, l'État doit cesser d'entraver les dynamiques locales et se recentrer sur ses missions régaliennes en outre 2023, déjà marqué par la suppression de 100 pour 100 de la taxe d'habitation pour nos concitoyens, l'État revient à la charge avec la suppression d'un autre impôt local la CVAE encore une fois, l'État choisi de supprimer un impôt qui ne lui appartient pas le lien qui unit les habitants et les professionnels d'un territoire avec le financement des services publics locaux, tu seras demain totalement rompu cela pour quel résultat : la taxe d'habitation a été supprimé, mais le pays n'a jamais connu autant d'impôts, nous venons de franchir les 45 % de prélèvements obligatoires, ce gouvernement fait payer une nouvelle fois aux collectivités locales, des choix unilatéraux qui seront lourdes de conséquences et permettez-nous de douter de la sincérité d'une compensation à l'euro près, qui n'a jamais été qu'un supplétif temporaire à la baisse des ressources des collectivités dans cette situation-là, la hausse de la DGF prévue pour 2023 est totalement insuffisante, rappelons que la DGF n'est pas un don mais un du qu'est-ce que cette hausse prévue de 330 millions d'euros face au 800 millions d'euros au bas mot, que l'inflation va coûter aux collectivités, cette année, au final, le prélèvement de l'État sera supérieur à ce qu'il était quand tu la DGF était gelé, enfin, comment ne pas faire allusion au retrait brutal de l'État au financement de l'apprentissage dans la fonction publique, qui porte un nouveau coup aux collectivités territoriales, il y a un an le gouvernement là Cnfpt et les employeurs territoriaux avaient trouvé un accord sur un mode de financement pérenne de l'apprentissage dans la fonction publique territoriale, par un amendement discrètement insérée dans le projet de loi de finances pour 2023, le gouvernement s'est clairement déclaré ne pas être disposé à tenir ses engagements, pourtant, il s'agissait d'un accord donnant-donnant dans lequel les collectivités ont accepté de payer une cotisation supplémentaire de 0 1 % de leur masse salariale en l'échange d'un financement du dispositif de soutien à l'apprentissage. Tous ces actes de défiance à l'égard des collectivités locales nuisent profondément à la confiance indispensable à toute relation et nous démontre une nouvelle fois un décalage criant entre les déclarations de bonnes intentions et les actes à l'égard de notre collectivité et pourtant, en cette nouvelle période de crise, il convient plus que jamais de soutenir les locomotives de notre pays et soyez-en les communes maire à leur tête en font partie, je vous remercie. Dans la suite de la discussion, la parole est à monsieur Max Brisson pour le groupe Les Républicains pour quatre minutes. minutes. Ce président, madame la ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, je ne suis pas un spécialiste des finances locales, à moins que le soit tous au Sénat, c'est donc avec mon coeur, même si je suis le dernier à m'exprimer, je vais dire ce que je ressens d'autant plus que je suis l'élu d'un département qui compte la plus grande intercommunalité de France avec 158 communes et 238 conseillers communautaires, Madame la Ministre, lorsqu'on parle de collectivités locales avec le gouvernement, les actes contredisent tellement les déclarations qu'on se demande si nous parlons la même langue, alors que le président de la République, annoncé son intention d'ouvrir un nouveau chapitre de la décentralisation vous présenter un projet de loi de finances, qui rétablit une forme de tutelle prolongeant l'esprit des contrats de Cahors, alors que le président République confirmé sa volonté décentralisatrice, vous réduisez les crédits de la mission à périmètre constant et quand les maires et l'ensemble des élus locaux crient leur détresse face à l'inflation et l'explosion des coûts de l'énergie, vous proposez un mécanisme dont comprend finalement qu'il ne va concerner que peu de communes et que ces critères son compte à peine compréhensible même pour les directions départementales des finances publiques, tout cela avant d'ouvrir la fois à sa modification permettez-moi donc de m'interroger sur la politique que vous engagez à l'écart des collectivités et pourtant et pourtant combien un nouvel acte de décentralisation serait nécessaire, combien la loi notre notamment qui rentre de grandir ta communalité a profondément bousculé l'exercice des responsabilités locales, 6 ans après, nous en supplie auront encore les travers et nous cherchons toujours en corriger les excès en attendant, les maires des petites communes, constate chaque jour qu'ils ont perdu la table Will compter pour participer à de grands des assemblées qui ne comprennent plus et à des commissions où dominent les jargons du moment ne serait il pas temps de remettre en cause sans remettre en cause le regroupement de 2016 de réfléchir à une meilleure territorialisation de l'action publique au sein des EPCI XXL, certains parlent de communes nouvelle n'est pourtant la résistance et là on ne peut pas non plus n'ignorait il faut peut-être réfléchir à des choses intermédiaires au moment où la proximité a montré toute son utilité lors de la crise de la Covid cas, c'est peu dire combien la montée en compétence des grandes communautés de communes, a dissous la voix des maires des petites communes de France, noyé dans de grands ensembles ils ne décide plus de mesures qu'ils auront pour qu'auront sur le quotidien des habitants qu'ils devront expliquer à des habitants qui ne manqueront jamais de leur demander des comptes, il faut donc leur apporter une réponse sous peine d'une terrible crise des vocations, la réduction de leur capacité à fixer le taux a également réduit leurs ressources fiscales et accru leur dépendance aux dotations et aux subventions désormais le pouvoir du maire se réduit trop souvent à demander et éventuellement obtenir des confidences mort pour les projets qu'il porte alors qu'il pouvait jadis engager la commune dans une politique de long terme et se donner ainsi plus de moyens pour tenir ses engagements et ne parlons pas des difficultés du temps considérable, passer à répondre à des demandes de plus en plus complexe, d'une administration entre souvent vertical éloigné qui les Corses dans des rapports, des normes et des procédures et pourtant et pourtant combien malgré la dépossession et l'aspiration des compétences demeure grande la vitalité communal, c'est oh con, maire de ce pays qu'il faut redonner des moyens du pouvoir et de l'espoir au contraire et à rebours de toute ambition décentralisatrice, ce budget à une matrice, il prolonge le démantèlement de la libre administration des collectivités et amplifient leur perte d'autonomie, il s'inscrit à long terme dans une logique, celle de la soumission des communes au bloc communal dans la droite ligne des dernières écritures de la Cour des comptes, il affaiblit dès à présent l'investissement local, au fond, il exclut toute relation de confiance et donc toute ambiance sereine, propice à nouvelle est indispensable, acte de décentralisation. Merci, cher collègue. La parole est à Madame Dominique Faure Ministre délégué chargé des collectivités territoriales et de la ruralité pour quinze minutes. Merci monsieur le président, messieurs les rapporteurs, mesdames et messieurs les sénateurs, notre gouvernement vous soumet aujourd'hui la mission Relations avec les collectivités territoriales RCT qui porte une partie de l'effort financier de l'État en faveur des collectivités, une nouvelle fois notre soutien sans faille aux élus locaux et aux territoires surtout face au défi inédit qu'ils doivent relever en ce moment avec l'inflation et la hausse du coût de l'énergie, c'est bien sûr une question de moyens, l'État est au rendez-vous avec l'ensemble des dispositifs d'aide d'urgence, le filet de sécurité, le bouclier tarifaire et l'amortisseur électrique pour un montant global de 2,5 milliards d'euros, mais également avec la hausse de 320 millions d'euros de la DGF inédite depuis 13 ans qui permettra la hausse ou le maintien de la dotation pour 95 % de nos communes, c'est également une question de méthode, notre gouvernement a construit ce projet de loi de finances, avec les associations d'élus dans une démarche de concertation sincère, c'est-à-dire une concertation qui a eu lieu, bien en amont, avec Christophe Béchu et Gabriel Attal, le gouvernement n'a cessé d'échanger avec elle tout du long, de l'élaboration de ce budget pour qu'ils répondent à leurs besoins, nous n'avons cessé d'être à l'écoute de les remontées du terrain comme de leurs propositions et le congrès des maires de France, a été un cadre précieux pour poursuivre ce dialogue essentiel preuve de sincérité de notre démarche, nous avons le souci de faire évoluer et d'affiner l'ensemble de ces mesures en fonction des retours des élus locaux et de l'évolution constatée de la situation dans nos territoires en témoigne notamment la révision de la hausse de la DGF passer de 210 millions envisagés initialement à 320 millions d'euros, la mise en place de l'amortisseur électrique pour compléter le bouclier tarifaire pour l'ensemble des communes qui ne sont pas éligible ou encore la volonté de simplifier les critères d'attribution du filet de sécurité et la modification du pacte de confiance que la première ministre a annoncé en clôture du congrès des maires, l'État s'engage résolument aux côtés des collectivités, des élus locaux et les dispositifs couverts par la mission RCT en témoigne avant d'entrer dans le détail des programmes 119 et 122 qui nous concerne aujourd'hui une vision d'ensemble de l'engagement de l'État aux collectivités, aux côtés des collectivités territoriales au sein de ce projet de loi de finances pour 2023 me semble nécessaire à périmètre constant, les concours financiers de l'État aux collectivités sont en hausse de 1,4 milliards d'euros par rapport à 2022, sans compter les amendements qui seront adoptés sur la mission notamment le complément de la compensation CVAE qui abondera le fond Vert, les 2 programmes de la mission RCT 119 et 122 représentent à eux 2 un peu plus de 8 % de ses concours financiers avec 4 milliards les concours financiers aux collectivités, qui regroupe les crédits de la mission, ainsi que les prélèvements sur recettes de l'État et certains transferts de TVA aux départements et régions pèseront E 43 milliards 897 millions d'euros en 2023, enfin l'ensemble des transferts financiers de l'État aux collectivités, lorsque l'on ajoute les dégrèvements et la fiscalité transférée s'élève à 107 milliards 700 82 millions d'euros, en hausse par rapport à 2022. La mission Relations avec les collectivités territoriales est composé comme vous le savez, du programme 119 et du programme 122 le programme 119 concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements inclus, d'une part, l'ensemble des dotations d'investissement par lesquels l'État accompagne les projets des territoires dans une logique d'effets de leviers et, d'autre part, l'ensemble des compensations des charges transférées aux collectivités dans le cadre de la décentralisation ou des pertes de produits fiscaux conséquentes à des réformes des impôts locaux, mise à part l'abondement exceptionnel de 303 millions d'euros de la dotation de soutien à l'investissement local a décide de l'an passé les autorisations d'engagement des dotations d'investissement DETR décile DPV décidé sont maintenues pour 2000 23 au même niveau qu'en 2022 : et si la décide exceptionnel n'est naturellement plus alimentés en autorisations d'engagement, c'était son côté exceptionnelles liées au plan de relance de 115 millions d'euros de crédits de paiement sont prévus en ouverture afin d'accompagner la réalisation des opérations lancées en 2020 et 2021, c'est autant de crédit qui allait monteront en plus la trésorerie des collectivités se sont ainsi un milliard 850 millions d'euros de dépenses d'intervention qui sont prévus en soutien au projet des communes et des groupements de communes et près de 212 millions d'euros prévue en soutien au projet des départements et des régions, l'ensemble des collectivités territoriales bénéficient ainsi d'un soutien stable et conséquent de l'État avec un puissant effet de levier financier au service de leurs projets sur le terrain, notons également la poursuite du plan Marseille en grand, elle a été cité, les 254 millions d'euros de tours d'autorisations d'engagement inscrit en 2022 ne sont naturellement pas reconduit dans le PLF 2023 mais nous prévoyons déjà 30 millions d'euros de décaissement dès l'année prochaine la même logique prévaut pour le plan d'action pour la Seine-Saint-Denis, pour lequel 10 millions d'euros de crédits de paiement sont prévues après les 20 millions d'euros engagés en 2022. La dotation Titres sécurisés la DTS, quant à elle, fait l'objet d'un effort inédit, avec une hausse de ses crédit de 20 millions d'euros permettant une hausse de sa part forfaitaire ainsi qu'une hausse de sa part incitative afin d'améliorer les performances des services concernés et résorber leur engorgement leur engorgement dommageable pour nos concitoyens, le développement de plateformes numériques permettra d'améliorer encore les délais de délivrance la dotation biodiversité est augmenté de 10,7 millions d'euros, cela correspond à une hausse de 44 % des moyens qui lui sont consacrés, pour 2023 pour atteindre un montant de 35 millions d'euros, ils avaient déjà été doublés en 2022 cette mesure apportent des moyens nouveaux aux communes classé parc national zone Natura 2000 où dorénavant aussi parc naturel régional le programme 122 Concours spécifiques et administration regroupe principalement des aides spécifiques alloués par l'État aux collectivités, confronté à des circonstances exceptionnelles, telles que des événements climatiques et géologiques de grande ampleur, son montant et stables en autorisations d'engagement est en hausse de 27 % en crédits de paiement, il témoigne de l'engagement continu de l'État aux côtés des collectivités fragilisées, en particulier face aux conséquences du réchauffement climatique, les suites de la tempête Alex mobilise d'importants moyens, tant pour la réparation des dégâts que pour le cadre du fonds de reconstruction un 1000000 d'euros d'aide sont spécifiquement débloqué pour les communes forestières, victime des scolytes face au défi financier inédit que connaissent les communes aujourd'hui l'enveloppe prévue pour les communes en grande difficulté financière et considérablement augmenter le montant des crédits nécessaires pour 2023 étant désormais fixé à 9 millions d'euros en autorisations d'engagement et en crédits de paiement, les collectivités d'outre-mer ne sont pas oubliés, la dotation globale de compensation, la DGSE de la Nouvelle-Calédonie, par exemple, est revalorisé à hauteur de l'inflation, enfin, nous avons à coeur, comme vous le savez, de favoriser la participation de toutes et tous à la vie politique de notre pays, en particulier au niveau local, le remboursement forfaitisée des frais de garde des élus mesure portées dans ce PLF et qui permettra d'améliorer sensiblement leur vie quotidienne, se traduit par la sortie du dispositif de remboursement du programme 122 et son inclusion dans la dotation particulière relative aux conditions d'exercice des mandats locaux la DP E L cette dotation sera maintenu à partir de 2023 pour les communes nouvelles qui vont se créer. Mesdames et messieurs les sénateurs, vous le voyez, la mission RCT marquée par la continuité de l'action de l'État pour accompagner toutes les collectivités locales à la fois dans les situations d'urgence, mais aussi dans leurs investissements de long terme, elles témoignent selon moi d'un projet de loi de finances solides qui répond aux besoins des collectivités avec le souci de n'en laisser aucune de côté, c'est à vous, désormais qu'il appartient de voter cette mission dans l'intérêt général de notre pays, de nos collectivités. Et de nos élus, un intérêt général qui n'est pas pour reprendre la définition de Rousseau, la somme des intérêts particuliers, mais bien l'intérêt des individus en tant que membre de la vie politique. Je pense que le PLF pour 2023 et la mission RCT en particulier constitue le bon équilibre entre soutien indispensable aux collectivités en ces temps difficiles en fonction de leurs besoins et la nécessaire poursuite collective de notre objectif de maîtrise de la dépense publique, j'espère sincèrement qu'un consensus peut se dégager dans cette assemblée sur cette mission à l'aune du dialogue constructif que nous avons mené ensemble et qui a conduit ce texte a évolué, cet esprit de compromis, cet esprit de consensus habite comme vous le savez, l'ensemble des assemblées locales, au-delà de toute logique partisane inspirons-nous toujours davantage de leur sens des responsabilités et de leur sagesse démocratique, je vous remercie. Merci madame la ministre, donc juste avant l'examen des amendements, je rappelle que que cette mission a une durée de d'examen de huit heures et que donc ça nous amènera à la fin de cet examen, à 20 heures ce soir,

Donc, nous commençons avec l'amendement 400 60 et 11 à l'article 27 monsieur Joly. Bonjour monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, mettre en place un programme village du futur de la même manière qu'il existe un programme Coeur de ville, qui concerne les villes de plus de 20000 habitants à un programme Petites Villes de demain qui on serre les deux à 20000 l'idée est de faire ainsi de donner les moyens au village nos village de 400 600000 1200 habitants qui offre des services de 100 alité à l'ensemble de la population des campagnes et qui donc participent au maillage de notre territoire, c'est une manière également symbolique de montrer à ces villages à ses habitants à aux élus qui les gère également que partie sont partie prenante de la France et et de son avenir et les proposer de demander à ce que la ministre lève le gage pour ce programme qui est évalué à 250 millions je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur. Oui, nous débutons effectivement par un amendement sympathique cet amendement néanmoins fait fait un peu double usage avec le peu de programme Petites Villes de demain, d'ailleurs, à titre personnel, ma commune qui a 700 habitants et Petites Villes de demain, donc ça rentre à l'intérieur et donc on je pense que ce serait créer un nouveau programme qui aurait finalement la la même cible, ce qui ne paraît pas une solution, même si il faut réfléchir sur la question pour ça que nous, la commission des finances ne peut être que défavorable. Merci ma ma Ministre. Merci monsieur le président, Mesdames et messieurs les sénateurs, la première ministre lors de sa déclaration de et Monsieur le Sénateur, joli, pardon, la première ministre lors de sa déclaration de politique générale à l'Assemblée nationale, a annoncé que le gouvernement mènerait prochainement un 2ème souffle de l'agenda rural afin de poursuivre l'accompagnement des territoires ruraux dans ce cadre et sous l'égide de la secrétaire d'État chargée de la ruralité, que j'étais 6 groupes de travail ont été mis en place au mois d'octobre 2022 sur des thématiques complémentaires à celles du Conseil national de la refondation et en complément des travaux qui vient d'être lancés sur la révision des zones de revitalisation rurale les conclusions de ces groupes de travail sont attendus pour la fin de l'année 2022, vous avez été, certains d'entre vous, largement associés je vous, vous vous en remercier viendront alimenter ce nouvel acte de l'agenda rural début 2023 parallèlement un travail d'évaluation du premier acte d'agenda rural a été confiée à Lee GE d'aider l'inspection générale de l'environnement et du développement durable, qui rendra ses conclusions à mi-janvier 2000 23 au regard de ce calendrier de travail, le gouvernement juge précoce, la création de nouveaux programmes à destination des territoires ruraux et vous demande donc le retrait de votre amendement. Merci monsieur Joly il est maintenu. Je le maintiens, monsieur le président, nous ne revendiquons pas lorsqu'on des représentants de ces villages, la qualification de ville et donc il est important effectivement qu'il y a un programme qui soit étiez à nos villages. Merci donc je mets voix le quatorze pardon Monsieur Delcros. Oui, merci Monsieur le Président, je je ne sais pas si ce PLF 2023 et et et le moment opportun pour pour pour voter cette idée, mais en tous les cas, je trouve l'idée tout à fait intéressante et et Madame la Ministre, je pense que il faut pousser jusqu'au bout la logique de l'accompagnement des territoires, il y a le programme Coeur de ville, ça a été dit ensuite le programme Petites Villes de demain qui s'adressent plutôt à on va dire des bourgs entre ancien chef-lieu de canton je trouve qu'il serait intéressant de pousser la stratégie d'accompagnement des territoires jusque dans la proximité des communes à travers un un programme qu'on peut appeler des villages d'avenir et je pense que le travail que vous menez pour donner une suite à l'agenda rural pourrait être l'occasion, en effet, de de réfléchir et et de porter ce programme en tous les cas, je pense que l'idée mérite vraiment une attention particulière. Merci, cher collègue, donc je mets aux voix l'amendement 471 avec 2 avis défavorables qui est pour.

Merci qui est contre. Qui s'abstient, il n'est pas adopté. 2 amendements en discussion commune le 643 madame Jospin. Merci monsieur le Président, c'est un amendement présenté par notre collègue, Annie ne le le oui ou qui concerne la revalorisation de 4 % des allocations concernant le RSA, il est nécessaire d'augmenter cette allocation dans la mesure où l'inflation est augmenté est augmenté de 6 % donc en effet la revalorisation du RSA à hauteur du niveau de l'inflation est nécessaire pour permettre aux allocataires de ne pas sombrer dans la précarité, face à la montée des prix des denrées alimentaires, de l'énergie, par ailleurs, il est nécessaire de compenser la dépense sociale supplémentaire très lourdes pour les Budgets des départements, le coût pour les finances des départements est considérable : 120 millions d'euros pour 2000 22 et 240 millions d'euros pour 2000 23 au titre du RSA, il est donc proposé par cet amendement de compenser le coût, le coût financier de la revalorisation du RSA à 4 % et de porter à la hauteur de l'inflation actuelle merci. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, en fait, il s'agit de prolonger le positif de compensation de la revue les risques de la revalorisation de 4 % du RSA donc au bénéfice des départements. Si monsieur rapporteur. mes chers collègues, donc il s'agit d'quasiment identique puisque l'homme portait sur 240 millions de de réactualisation d'augmentation de revalorisation et l'autre sur 244 millions ce qu'on peut simplement dire à ce stade, c'est qu'en première partie, le Sénat a déjà indiqué votez un montant d'augmentation du RSA de 240 millions d'euros de compensation de 240 millions d'euros, donc ça a déjà été voté en première partie, donc c'est amendements sont satisfaits de ce point de vue là en admettant même que grade millions ne prospère pas ah au final il ne prospère aurait pas plus en première partie, comme 2ème partie donc je vous demande de de retirer ces deux amendements puisqu'ils sont déjà satisfaits merci. Merci madame la Ministre. Merci monsieur le président, hein, mesdames et messieurs les sénateurs, Madame Annie Le Houerou, dans un contexte de fortes hausses de prix, la revalorisation anticipée du RSA de 4 % a été votée par le législateur, par la loi, pouvoir d'achat pour anticiper l'augmentation annuelle du RSA sur l'inflation acté en avril de chaque année, cette mesure a déjà été accompagné d'un fonds de 120 millions d'euros pour les départements au titre de 2022 malgré l'absence d'obligation juridique de compensation, ce soutien se justifier par le fait que les départements ne pouvait pas anticiper cette revalidation revalorisation décidée par le gouvernement en dehors du dispositif habituel de revalorisation annuelle votre amendement propose de reconduire ce dispositif exceptionnel au titre de l'année 2023 et de le porter à 240 millions d'euros, nous y sommes défavorables pour plusieurs raisons : premier le, le Sénat a déjà voté une telle compensation en première partie du PLF, contre l'avis du gouvernement, ça vient d'être dit par ailleurs une telle compensation ne se justifie pas, alors qu'il était établi que les dépenses 2021 de RSA sont en baisse par rapport aux dépenses de 2020 et que les dépenses de 2022 suive cette même tendance, enfin, je tiens à souligner que les départements bénéficient par ailleurs de ressources fiscales très dynamique, les droits de mutation à titre onéreux, la TVA qui peuvent contribuer au financement de leur politique d'insertion, les DMTO pourrait se maintenir en 2022 au niveau exceptionnel de 2021 et la dynamique de TVA des départements atteindra 9 6 % en 2022, et pourrait atteindre plus de 5 % 2023 en conséquence le gouvernement vous demande le retrait de cet amendement, sinon il est défavorable, merci. Si Madame Jospin, il est maintenu.

Qui est contre qui s'abstient, il n'est pas adopté cet amendement discussion commune de 449 monsieur Sautarel. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, en fait, cet amendement vise à créer un un nouveau fonds destinés aux travaux de voirie communale pour les communes de moins de 500 habitants qui pourrait aussi bien s'inscrit dans le prolongement de l'agenda rural mais aussi répondre au au souci de mobilité durable qui nécessiteront quoi qu'il en soit, ce sont des territoires ruraux, le maintien d'infrastructures routières, il existe en effet un 1000000 de kilomètres de voies communales dans les 1000 17000 communes de moins de 500 habitants qui, aujourd'hui, je l'ai rappelé aussi dans la discussion générale, tout à l'heure sont un des points de charge les plus conséquents pour ces communes et en même temps les plus inégaux puisque ils ne sont pas en lien Direct avec la population, mais avec la longueur de voiries existantes sur ces communes en conséquence la la proposition que je fais à travers cet amendement de créer ce fonds en en ponctionnant des crédits sur le programme, dont nous parlons et sur le programme 122 consisterait à établir un forfait kilométrique de 200 euros pour ces communes en terme de voirie communale de façon à prendre en charge une partie de ses charges très conséquente et qui souvent bloque tout autre investissement en conséquence, cet amendement vise à créer un fonds de l'de 200 millions d'euros, je vous remercie. Merci le quatre 400 cinq Madame Préville. Merci monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, cet amendement vise à augmenter la dotation de soutien à l'investissement local a et la dotation d'équipement des territoires ruraux, la DETR à la hauteur de 3 milliards d'euros afin de soutenir l'action des collectivités territoriales face à la crise énergétique et dans leurs objectifs pour la transition écologique, cet amendement propose une hausse à 100 millions d'euros, la situation des collectivités s'aggrave depuis des années, nous l'avons tous dit : il est urgent de mettre en place un soutien pérenne, face à une situation structurellement complexe pour les collectivités, elles font face à de nouvelles dépenses dues aux nouvelles compétences, notamment en matière de transition écologique et sociale, que ce soit pour la mise pour la mise en oeuvre des CRT RTE l'atteinte des objectifs climat-énergie de la France ou encore le 0 artificialisation nette avec son 1er palier de réduction de consommation d'espace en 2030 d'autant plus que les décrets qui sont pris sur ce sujet sont particulièrement difficiles à respecter et mettre en oeuvre, vous rendez compte 50 % d'ici 2030, c'est-à-dire en 8 ans seulement, alors que jusqu'à présent si peu a été fait et il y a une espèce de brutalité dans l'application de Cezanne, l'urgence climatique et sociale et là, mais les financements étatiques ne suivent pas cette réalité et tantôt stagne, tantôt diminue, or sans financement adéquat, tous ces objectifs, resteront à l'état d'intention et ne seront jamais traduit sur le je vous remercie. des personnes sans domicile stable par les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale C'est président madame la Ministre cet cet amendement concerne la dotation aux communes pour la protection de la biodiversité et la valorisation des militer rural j'en profite pour dire que la création de cette dotation a été une belle avancée en direction des territoires ruraux et une juste reconnaissance de l'apport qu'ils font à la société toute entière en matière de protection de l'environnement, elle a été la bienvenue, alors elle a été cette dotation élargi à l'Assemblée nationale et nous prévoyons dans des amendements futurs aussi un élargissement supplémentaire à la fois par rapport aux critères potentiel financier pour les parcs régionaux pour que les communes qui ont signé la charte d'un parc national puisse être éligible à cette dotation, ce qui n'était pas le cas auparavant, et puis nous fixe nous proposant de fixer un seuil minimum afin que ces évolutions positives que nous soutenons, bien entendu, en faveur des communes ne se traduisent pas par une baisse

Oui, merci Monsieur le le président, cet amendement vise donc à compléter les dispositions prévues à l'article 46 du projet de loi de finance, un dispositif qui prévoit une distinction entre les communes situées dans le coeur d'un parc national et les autres communes du parc, or il semble que cette distinction ne soit pas pertinente, d'autant que chacune et signataire de la charte du parc national aussi cet amendement qui avait été également porté par Joël Giraud ancien Ministre de la ruralité prévoit en particulier l'extension de l'éligibilité de la infraction parcs nationaux de la dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité et pour la valorisation des aménité rural cette extension bénéficierait donc aux communes dont le territoire est situé en tout ou partie dans un parc national mais hors zone de coeur merci. amendement propose d'instituer une dotation aux communes non éligibles à la compensation de la taxe sur les spectacles, en dépit des investissements, un équipement sportif qu'elles ont engagées peut avoir la suppression en 2015 de la dite taxe pour les manifestations sportives, en 2015, le texte a prévu de ne plus soumettre à la taxe communale sur les spectacles, les droits d'entrée perçus par les organisateurs des manifestations sportives, mais en parallèle, un prélèvement sur les recettes de l'État avait été institué pour compenser les pertes des recettes, suivie par les dites communes, d'un montant égal au produit reçu en 2013 ce dispositif n'avait cependant pas tenu compte de la situation de communes qui bien que ne percevons pas la taxe sur les spectacles otite des manifestations sportives en 2013, par conséquent, ne éligible au PSR de compensation s'était elle-même engagé dans des projets d'investissements en équipements sportifs de grande ampleur et compter précisément sur ces recettes pour assurer la charge financière qu'elle devait prendre en compte, lié à l'équipement pour objet de combler cette lacune en instituant une dotation qui serait versée aux communes ayant commencé au plus tard le 1er janvier 2014 la construction d'un nouvel ouvrage destiné à accueillir des manifestations sportives pouvant recevoir plus de 5000 personnes, son montant sera égal à 8 % du montant des recettes brutes de manifestations sportives organisées dans l'enceinte de l'eau du dit ouvrage au cours de la première année durant laquelle l'ouvrage je vous fais grâce a fait l'objet d'une exploitation ce taux correspond en fait au tarif de droit commun à appliquer avant la suppression de la taxe, c'est une un rééquilibrage qui me paraît utile, nécessaire, je vous fais grâce explication purement financière, sur lequel s'appuie cet amendement et dont il est évidemment tenu compte dans celui-ci, merci. monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, alors là le l'objet de cet amendement d'appel et d'abonder les crédits dédiés à la dotation de soutien à l'investissement local pour donner les moyens financiers nécessaires aux collectivités territoriales d'assurer la transition énergétique tout en réduisant leurs charges courantes, le rapport publié en juillet 2022 par la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation du Sénat portant sur la hausse du coût des énergies et son impact pour les collectivités territoriales établi que, depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, la facture énergétique des collectivités territoriales explose les dépenses énergétiques oh mon Dieu, 50 pour 100 dans les petites villes et varie jusqu'à 300 % pour certaines communes et un peu plus dans les communes touristiques cette se met en péril des services publics locaux essentiels et porte le risque d'un roman le chemin des collectivités à leurs projets d'investissement dans ce contexte international et afin de donner les les capacités aux collectivités locales de réduire leurs charges courantes et de participer à la réduction de gaz à effet de serre, je vous propose de renforcer les capacités d'investissement public local orienter spécifiquement vers la transition écologique pour recentrer les crédits accordés à la mise en oeuvre et la transition énergétique Madame la Ministre, vous allez certainement me répondre : à quoi bon augmenter les les crédits d'un Fonds dans l'enveloppe n'est pas consommées chaque année, pourquoi je pense qu'il faut se poser la question parce que, d'après les maires là des il est très compliqué à mobiliser, à la différence de la DETR certaines un particulier dans les petites communes ignorent même que ce dispositif existe alors, à défaut d'augmenter l'enveloppe des crédits des îles de grâce : faites en sorte de simplifier les procédures d'accès à ce fonds, merci, merci, chers collègues, monsieur le rapporteur. Bon, je vais essayer de répondre aux cet amendement un peu différente dans leurs objets, alors tout d'abord, l'amendement 449 pour la création d'un nouveau programme, doté de 200 millions d'euros destinés aux travaux de voirie communale pour les communes de moins de 500 habitants, alors c'est un sujet indiscutablement sérieux, c'est un problème dans quelques, dans les territoires sur le financement de ces travaux de voirie, je voudrais simplement dire d'une part, il y a sans doute un problème de de calibrage de l'amendement parce que demander de 100 millions d'euros, en gros, c'est demander pour bien à peu près un tiers à 40 % de la déciles national, donc il s'agit vraiment d'une enveloppe, vous ouvrez la porte, si j'ai pu dire large chers collègues et donc je suis pas sûr que que le gouvernement, mais ils sont à nous le dire vous suivent sur ce montant on peut répondre de différentes façons, qui ne sont pas toutes satisfaisantes, mais qui s'ajoutent bien sûr les communes bénéficient du remboursement du FCTVA sur ses travaux sur tous les réseaux de voirie, bien sûr, elles peuvent bénéficier de la DETR ou de la décident, mais en réalité, on sait que ce sont des enveloppes sur lequel il est difficile aujourd'hui d'imprimer de la voirie et donc on est, on est conscient que ce sont des réponses finalement point point par point, département par département, qui permet éventuellement de de prendre dans la DETR, ce type de de dépenses et, enfin, il faut toutefois pas oublier un partenaire qui peuvent soutenir ces travaux qui sont les évidemment les les départements au titre de l'aide aux communes, là aussi, les soutiens sont variables d'un département à l'autre, mais ça reste des solutions et donc, nous serions plus tôt pour considérer, vu le montant qu'il s'agit d'un amendement d'appel et et que le gouvernement nous répondent et vous proposez en tant que commission un retrait. le quatre cent cinq donc, qui vise à augmenter de 100 millions d'euros, les crédits de la DETR dès la déciles afin de soutenir l'action des collectivités territoriales face à la crise énergétique. Donc évidemment, je crois que dans cette assemblée, tout le monde partage la préoccupation la question évidemment, c'est de trouver la la bonne solution, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a quand même un certain nombre de dispositifs qui sont maintenant prévues d'abord effectivement l'amortisseur sur l'électricité qui devrait permettre de réduire la hausse de la facture énergétique qui représentent des montants très significatifs, deuxièmement quand cet amortisseur n'est pas suffisant, il sera complété par le filet de sécurité qui prendra aussi en charge d'une partie de la hausse des dépenses énergétiques, et par ailleurs la décide rénovation énergétique comme le font friche et le Fonds renaturation des friches permettent déjà aux collectivités d'engager des travaux dans ce sens et puis il reste mais je reconnais qu'on est encore un peu dans le flou, l'enveloppe fond Vert qui pour une partie pourrait certainement venir donc la Commission considère en tout cas que si la question est juste, il y a déjà beaucoup de, de, de, de solutions qui sont apportées, en tout cas dans les principes, par le gouvernement pour répondre à ces enjeux et besoins dans ce domaine et que donc il faudrait au moins attendre d'avoir un retour sur ce qui se fait avec ses investissements et ses moyens pour éventuellement abondé ces enveloppes donc plutôt une demande de retrait concernant l'amendement 645 qui vise à ouvrir 10 millions d'euros supplémentaires aux communes, pour financer les dépenses liées à l'activité de domiciliation des personnes sans domicile stable par les Centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, nous considérons que nous n'avons pas de données de données consolidées sur l'ensemble du territoire et que les rapports ne sont pas toujours accessibles en ligne, si bien que nous manquons d'informations pour mesurer la charge de cette activité et son coût pour la collectivité et donc nous demandons l'avis du gouvernement concernant l'amendement 98 rectifié cet amendement majeur, les crédits de la dotation de biodiversité de 7,3 millions d'euros sur ce montant 6,7 millions d'euros doivent permettre le versement d'un montant minimum de 3000 euros à chaque collectivité bénéficiaire, quelle que soit la fraction contre 1000 euros actuellement, l'objectif est, en effet, et que le minimum perçu, soit le même pour toutes les fractions alors que jours il est fixé, fixé à 1000 euros pour les par Natura 2000 parcs naturels régionaux et parcs marins alors qu'elle est de 3000 pour la fraction parcs nationaux, il y a donc une volonté d'un traitement égal des communes qui réalise des dépenses liées à la protection de la biodiversité, nous vous proposons un avis de sagesse concernant l'amendement 400 de de madame cet amendement major également les crédits de biodiversité de 4 millions d'euros, il fait donc le même objet que l'amendement 98 mais avec un chiffrage inférieur et je demande donc sort son retrait au profit de l'amendement 98 qui est chiffré à 7,3 millions d'euros. Concernant maintenant l'amendement 698 du président buffet le présent amendement propose d'instituer une dotation aux communes non éligibles à la compensation de la taxe sur les spectacles, en dépit des investissements, un équipement sportif qu'elles ont engagées peut avoir la suppression en 2015 de la dite taxe pour les manifestations sportives, donc si les effets cliquez qu'on connaît bien, quand une loi s'applique avec des possibilités de pertes dans le dispositif de compensation sur la base du produit perçu en 2013 ne tient pas compte de la situation des communes qui s'était engagé dans des projets d'investissement avant même que la loi de Pass donc opposition sagesse pour le je crois que c'est le dernier l'amendement numéro 557 il a été indiqué que c'était un amendement d'appel donc la même réponse vaut sur le fait qu'il y a effectivement des outils qui sont mis en en oeuvre et qui doivent qui doivent permettre de financer les collectivités territoriales pour la transition énergétique et écologique, sans doute pas dans les moyens suffisants, mais mettons-les en oeuvre avant d'aller plus loin, qui plus est demandé un 1000000 d'euros, c'est très raisonnable chère collègue et donc ça ramène bien un amendement d'appel dont retrait si vous le voulez bien. Merci, monsieur le rapporteur, Madame la Ministre. Merci monsieur le président, Mesdames et messieurs les sénateurs, je vais essayer d'être aussi concis ce que monsieur le rapporteur, concernant le 449 vous proposer la création d'un fonds de 200 millions d'euros destinés aux travaux de voirie communale pour les communes de moins de 500 habitants pour les mêmes raisons que monsieur le rapporteur, et pour ne pas vous relire ce que je vous ai dit dans mes propos liminaire, je vous invite à retirer cet amendement, sinon l'avis du Gouvernement sera défavorable.

vous proposer d'instaurer un abondement de la dotation de soutien à l'investissement local a déciles et la dotation d'équipement des territoires ruraux, la DETR de 100 millions d'euros en 2022 pour les mêmes raisons que l'amendement précédent, nous vous demandons le retrait, comme monsieur le rapporteur, sinon dans la position du Gouvernement sera défavorable. L'amendement 645 présenté par la sénatrice Michèle Meunier. L'obligation légale de domiciliation, prévu par la loi Dalo du 5 mars 2007 lorsqu'elle est exercée de manière facultative par les CCAS ne constitue pas un transfert de compétences au sein au sens de l'article 72 tiré de de la constitution, elle ne nécessite donc pas une compensation depuis 2017, le montant des concours financier stable, les communes disposent bien des moyens nécessaires. Pour financer les CCAS, sans qu'il soit nécessaire de mettre en place une nouvelle dotation l'augmentation de la DGF ne rempliraient pas l'objectif de l'amendement, car les modalités de répartition de cette hausse ne sont pas définies en outre cette loi de finances prévoit un ensemble de mesures de soutien budgétaire en faveur des collectivités locales, notamment comme je l'ai déjà dit plutôt pour leur permettre de faire face à l'inflation, pour n'en citer qu'une : pour la première fois, puis 13 ans, la dotation de globale de fonctionnement est augmenté de 320 millions d'euros par des crédits nouveaux de l'État pour l'ensemble de ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable. Pour ce qui est de l'amendement 557 présenté par Monsieur. De 98. Nous sommes d'abord en 98 là.

Vous proposez de majorer les crédits de la dotation biodiversité et aménité rural à hauteur de 7 3 millions d'euros pour un transfert du programme 122 vers le programme 119 les majorations compenserait effectivement les coûts des mesures proposées afin que les communes déjà bénéficiaires de la dotation ne subissent pas une baisse de leur attribution au au regard de l'application d'un montant minimum de 3000 euros pour chaque fraction et de l'élargissement du périmètre d'éligibilité de la fraction parcs nationaux, en revanche, ces crédits ne pourrait pas être prélevés sur l'action, hein, du programme 122 qui ont vocation à financer des aides exceptionnelles de l'État aux collectivités territoriales, au regard de ces propositions qui vont dans le sens d'un verdissement renforcé des concours financiers de l'État aux collectivités tout en évitant des effets de bord préjudiciable pour les communes déjà bénéficiaires de la dotation, je m'en remets je crois comme monsieur le rapporteur à la sagesse de votre assemblée. L'amendement 402 qui est présenté par la sénatrice Nathalie Delattre, vous proposez d'abonder les crédits du programme 119 de 4 virgule 1 millions d'euros pour 600000 euros afin de compenser l'élargissement aux communes, or, coeur de parc national et pour 3 5 millions d'euros fait financer le relèvement du montant minimum global d'attribution individuelle aux communes pour le fixer ah. Trois mille trois

composant la dotation, dès lors, cela impliquerait de déterminer sur quelle fraction porterait le relèvement du seuil ou de relever le plancher de chaque fraction qui est actuellement de 1000 euros avec un abondement supplémentaire pour neutraliser le coût de la mesure, c'est ce que fait l'amendement numéro 5 ans du sénateur Delcros, qui propose en outre une majoration supérieure des crédits de la dotation. Comme précédemment, et comme vous m'y avait invité, je vous demande madame la sénatrice le retrait de cet amendement. C'est l'amendement 698 qui est présenté par le sénateur François Noël Buffet l'article 21 de la loi du 29 décembre 2014 finances pour 2015 instituts un prélèvement sur les recettes de l'État, destinée à compenser les pertes de recettes pour les communes résultant de la suppression de l'impôt sur les spectacles, sur les droits d'entrée perçus par les organisateurs de manifestations sportives, la compensation est calculé en référence aux produits d'impôt sur les spectacles perçus sur ces manifestations sportives en 2013, s'il n'a aucune obligation en la matière, l'État compense la suppression des impôts locaux, décidée par le législateur, le plus souvent référence un produit historique effectivement perçu de la recette supprimer pour autant, il ne paraît pas possible de compenser une recette qui aurait été perçu si l'impôt n'avait pas été supprimé, ce qui est proposé en l'espèce, monsieur le sénateur par votre amendement en effet celui-ci crée une dotation afin de compenser la perte de recettes de taxe de spectacle qui aurait été générée par des investissements sur des équipements sportifs si la taxe n'avait pas été supprimé je le gouvernement vous propose une position défavorable. L'amendement 557 présentée par le sénateur Sébastien Pla c'est abondé la décide de millions d'euros supplémentaires, vous proposez de. Renforcer les capacités d'investissement public local orienté vers la transition écologique en abondant la déciles je vais pas rappeler ce que j'ai dit en propos liminaire, je vais pas rappeler ce qui a été dit de nombreuses fois rappeler ce fond Vert pour 2 milliards d'euros en 2023 la position du gouvernement est défavorable. Si Monsieur le Président, madame la miss, mes chers collègues, une explication de vote sur cet amendement, qui effectivement vise tous a abondé davantage de l'aide aux collectivités, même si ce sont même si cela se passe sur des sujets différents, nous les voterons s'ils sont maintenus, je, je tenais à attirer l'attention sur le premier amendement en discussion commune, celui de notre collègue Sautarel, parce qu'effectivement, nous avons aujourd'hui pour ces communes qui ont pourtant un nombre de de kilomètres de voirie. Extrêmement important, aucune autre aide possible pour pouvoir aménager et entretenir, à une époque, y compris où les engins agricoles d'aujourd'hui ne sont pas ceux d'il y a quelques décennies et donc donc des impacts sur ces voiries bien plus important précédemment, et à une époque aussi où pour un certain nombre de petites communes et je pense dans mon département, aux communes du Pays d'Urfé qui sont en bordure d'autoroute qui font que, systématiquement, aujourd'hui quand il y a des travaux des accidents, des fermetures de de Dax plus principaux les applications en tous genres, invite, y compris les poids lourds qui traversent notre pays de part et d'autre, à prendre des des chemins et à passer sur des voies Hucknall qui ne sont pas du tout adapté à ce type de trafic et qui viennent défoncer un peu plus encore la route et ajouté de coûts supplémentaires à ces petites communes pour assurer tout de même la continuité des déplacements, donc si notre collègue le maintien, nous nous le voterons un dernier mot pour finir parce que j'ai beaucoup entendu dans les arguments tendent la commission que de la ministre : un coup, ce n'est pas assez, un coup c'est trop une autre fois, ce n'est pas bien engagée, je rappellerai à chacun, ici, que vous êtes libre, madame et et monsieur de pouvoir sous-amender, vous êtes libre, y compris parfois de pouvoir lever les gages et que je crois que nous sommes là, avant tout, non pas pour faire de la gestion, mais pour faire de la bonne politique au service des collectivités territoriales de notre pays et donc les arbitrages de comptabilité qui sont fondamentaux, il vous appartient de pouvoir y répondre puisque vous en avez les pouvoirs alors que nous, en tant que petit parlementaire nous n'avons pas les pouvoirs. 449 de notre collègue Sautarel certes, monsieur le président de la commission des finances, on y va pas avec le dos de la cuillère 200 millions, un tiers de la décile et à titre personnel, je considère plutôt cet amendement que je vais voter comme un amendement d'appel parce que c'est vrai que les considérations de de l'exposé des motifs et et tout à fait clair, il est juste pas possible que on ne prennent pas en compte les besoins exprimés et qui ne sont malheureusement pas satisfait, comme on l'aurait souhaité par la DETR, mais également par un certain nombre de conseils départementaux qui n'interviennent pas, vous l'avez dit, monsieur le président de la commission des finances, on ne peut pas comme ça, ne pas tenir compte de tous ces besoins concernant les les les voies communales dont on le sait, hein, une grande partie ne sont pas toujours en bon état, tout particulièrement dans les communes rurales, la question que je me posais moi, elle concerne Monsieur Sautarel pourquoi 200 euros par kilomètre et nul doute que que, chers collègues, vous avez dû prendre quelque part, une référence en la matière, mais ces deux cents euros effectivement viennent considérablement si on le multiplie par le nombre de kilomètres concernés dopé la somme en question moi franchement je souhaiterais avoir plus d'informations sur le coût véritable occasionnée par ce type de travaux et à destination de Madame la Ministre, si on pouvait faire le clair en la matière, voir ce que ça coûte véritablement à tout le moins, encore une fois, en qualité d'amendements d'appel faire le le point sur cette situation, vous l'avez compris c'est tout à fait important pour les les collectivités concernées, enfin moi je le voterai au moins cet amendement qualité d'appel. Merci, oui merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, effectivement, quelques éléments de réponse par rapport à à cet amendement qui est, qui est un amendement de ou de sensibilisation, bien sûr, mais qui se veut aussi raisonnables, même si la somme peut paraître conséquente, je veux juste rappeler en remerciant le le président de la commission des finances, rapporteur spécial pour les arguments qu'il a développé, que je peux partager mais mais aujourd'hui je on on ne peut pas comparer ou en tout cas, se mettre en rapport sur cette enveloppe avec la décide, parce que la décide d'interdire absolument pas sur ces types d'investissement c'est aujourd'hui même difficiles parfois de le faire admettre dans le financement de la DETR, on se bat chaque année avec les collègues pour le faire prendre en compte et je suis de ce point de vue-là un peu inquiet sur les critères qui veulent être introduit de, de, de, de caractéristiques, même si elles seront facultatives de de verdissement des investissements éligibles à la DETR pour faire continuer à financer nos nos voiries nous voir communales, donc ça c'est, c'est déjà une une difficulté ensuite la libre administration des des départements, fait que les réponses sont hétérogènes sur le, sur le territoire, quant au calibrage du fond, c'est, c'est effectivement un calibrage aujourd'hui qui qui se voudrait un premier appel, hein, un 1er pas dans l'attendent sans doute d'une approche qui pourrait être affiné et qui répond aussi non seulement à tout ce qui a été dit en termes de charges et et en terme d'usage par des engins aujourd'hui de plus gros calibre, voire de voies de délestage qui sont aujourd'hui à la charge de des communes, mais aussi pour insister sur le fait que la mobilité dans nos territoires du roi avec des véhicules à moteur, que ce soit les automobiles ou d'autres types de de véhicules et que donc il est nécessaire d'entretenir ce maillage qui est, qui est riche et fort dans notre dans je, je regrette que Madame la Ministre n'est n'est n'est pas proposé d'examiner plus au fond, cet amendement pour apporter, peut être une réponse dans la durée, a un besoin qui est réel et il y a des communes qui se sentent abandonnés sur les chargements. Merci, merci, donc il est maintenu, la présidente de la.

mais figurez-vous que je ne vais pas le retirer parce que, avec l'accord de Bernard Delcros, s'il le veut bien, je le rends identique puisqu'il a trouvé la petite astuce financière mais donc je le rends identique, donc il sera maintenu dans cette condition est-ce que vous pouvez, du coup nous rappeler puisqu'elle tous les sujets sont intéressants si il y a d'autres amendements qui sont votés et qui font tomber les autres parce qu'on est en discussion commune ce qu'il n'y avait que le mien, qui maintenant est rendu identique qui souffrait cette règle merci. oui monsieur le président, j'aurais pu le dire mais bon. Oui je je voudrais d'abord vous dire que sur l'esprit, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, il y a pas difficulté par rapport au sujet routes communales des communes de moins de 500 habitants, il y a pas de sujet, on nous a rappelé que c'était un amendement d'appel, c'est ce que nous avons considéré, c'était un un mandat pas mon Open, alors pourquoi nous appelant au retrait, on comprend bien qu'il peut être votée il y a pas de problème, laisser dans la navette bon et on sait qu'il ressortira pas mais c'est pas grave, ça peut être une façon d'insister sur le sujet auprès de la ministre et nous le comprenons tous, pas de sujet, mais un petit problème, c'est que si on le met au vote, il fait tomber ce pour lequel nous avons une position de sagesse et positives donc et je, je, je vous le dis d'autant plus que ça nous est déjà arrivé la première fois que j'étais président de de présidents de commission, on a voté un premier amendement, vous vous en souvenez, pour les outre-mer un amendement de 5 milliards qui a, qui a tout dévasté, il a fallu qu'on s'arrête pour essayer de retrouver dégage pour les autres amendements et donc là les autres amendements ne serait plus gager et donc n'étant plus gager il tomberait donc voilà je, je pense qu'on peut partager tous l'idée qui est développée par cet amendement la gentillesse correction par rapport à vos collègues de ne pas le voter mais de dire le travail est fait, hé bien ça ne ferait pas tomber les autres, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci monsieur le président, c'est précisé donc. Monsieur Marie. Merci monsieur le président, je voulais revenir sur l'amendement 645 présentée par Madame Meunier et notre groupe pour rappeler que la Fondation Abbé Pierre, recense plus de 300000 personnes sans domicile en France et et que ce chiffre a doublé depuis 2012 et qu'il est important et impératif même de garantir leur accès au droit, à ces personnes, or ils éprouvent de plus en plus de difficultés à accéder au service municipal de domiciliation du fait de la saturation d'un certain nombre de CCAS qui manque malheureusement de de financement et et la domiciliation est devenu un droit opposable à la suite de la loi Dalo et ce droit a été renforcée par la loi, allure et une divergence avec Madame la Ministre, cette nouvelle obligation légale de domicilier n'a pas été de compensation financière, alors que c'est effectivement une nouvelle compétence et qu'elle relève donc de l'article 72 de la Constitution nous proposons donc une dotation complémentaire et j'ajoute que cet amendement est issu, proposition d'un collectif qui réunit Emmaüs, le collectif national des droits de l'homme, la Fédération des acteurs de la Solidarité, le Secours catholique Caritas France et soutenu par l'Union nationale des centres d'action sociale

de cet amendement pour appeler à Madame la Ministre, l'inquiétude des maires que nous avons rencontré un autre département, il n'y a pas si longtemps que ça, nous étions en présence tous les deux sur les difficultés d'accès que rencontrent les maires et leurs collaborateurs à l'accès à ces différents fonds que nous mettons en oeuvre régulièrement chaque année, donc cette jungle, ils sont complètement perdus aujourd'hui, moi je vous demande très sincèrement de simplifier les démarches et l'accessibilité à l'ensemble de ces fonds car la plupart de nos mères et en particulier ceux des plus petites communes ont l'impression de ne pas être alors nous pouvons débattre des heures et des heures à proposer des dispositifs inventer les trucs mais si, au final ça ne touche pas la cible et les communes qui en ont besoin, ça fonctionne pas et c'est dommage tout ce temps perdu cet argent pour rien, merci madame Louise. donc je vais mettre aux voix les amendements, il est retiré, monsieur souterraine. Par sagesse, je le retire, considérant que l'amendement a été entendu et par solidarité avec mes collègues, merci. Merci donc le 449 et retiré

Qui s'abstient, il n'est pas adopté le même vote pour 645. Même vote il n'est pas adopté, je vais, on voit le 98 et le 400 de qui est devenu identique avec un avis de sagesse de la commission elle sagesse du gouvernement qui est pour. Qui est contre qui s'abstient ils sont adoptés je mais au moins 698 avec un avis de sagesse de la commission, un avis défavorable du gouvernement qui est pour. Qui est contre qui s'abstient, il est à adopter et le 57 et retiré le 458 monsieur Bena Roche. Oui merci, excusez-moi, cet amendement a pour but de créer un fonds actions énergie climat pour permettre aux collectivités territoriales, de financer la rénovation de leur Pack de bâtiments scolaires, il faut savoir qu'en France les bâtiments représentent à peu près quarante-quatre % de nos consommations d'énergie finale un quart de nos émissions de dioxyde de carbone que près du trois quart du parc de bâtiments publics sont détenus par des collectivités territoriales et que les écoles, collèges et lycées comptent pour près de la moitié des surfaces, ce qui constitue bien entendu un coût important pour les collectivités, la réduction immédiate de la consommation d'énergie des bâtiments et donc une priorité pour permettre aux collectivités de moi des potes du coût des énergies fossiles et de diminuer leurs émissions de CO2, mais aussi pour permettre de dégager des marges de manoeuvre budgétaires alors que leurs finances affecté durablement par l'inflation, il faudrait pour cela engager des travaux immédiats pour moderniser l'éclairage, les menuiseries extérieures, remplacer les chaudières au fioul isolé les parois améliorer la régulation et la programmation des installations, ce qui peut permet également d'introduire des sources d'énergie renouvelables situations qui peuvent aller jusqu'à la mise en place de pompes à chaleur R O ou géothermiques ou à celle de capteurs solaires thermiques ou photovoltaïques sur les toits, ainsi que des chaufferies bois les dispositifs existants ne permettent pas de remplir efficacement cet objectif, les collectivités, faut remonter un éclatement trop important des sources de financement, et par ailleurs la part allouée à la rénovation au c'est au c'est des dotations d'investissement est souvent faible, la solution la plus efficace, nous semble donc être la création de fonds Haddock qui pourrait d'ailleurs être pilotée par la avec pour objectif de mieux répartir les demandes de rénovation des bâtiments scolaires, selon un plan pluri-annuel pour reprendre une suggestion du rapport remis au gouvernement en 2020 par François de Marc les préfets devrait pouvoir s'appuyer sur les directions départementales des territoires et sur les directions régionales de l'Ademe et la et de la CMA là où ce serait possible dès lors le présent amendement procède d'une part la création d'un nouveau programme sein de la mission intitulée Action énergie climat pour les bâtiments scolaires, crédité d'un montant de 20 millions d'euros et pour respecter les règles de recevabilité financière, une baisse de même montant de 20 milliards sur de 20 millions au niveau de l'action 01. Oui, mes chers collègues et chers collègues ben Roche il y a, il y a évidemment pas par rapport à l'exposé des motifs, la moindre difficulté par rapport à l'exposé des motifs, simplement le moyen utilisé, c'est-à-dire créer un fonds spécifique de 20 millions d'euros, qui finalement n'est pas un fonds d'ailleurs très importante étant fait couvert largement par les fonds disponibles et font classiques que soit la DETR, sur lequel il est clairement identifié, que ce type de projet doit doit s'inscrire, même sur la décide, classique, sans parler de la rénovation énergétique est maintenant totalement engagé et et puis bon ben là j'y vais avec beaucoup de prudence sur le fond Vert

Merci monsieur le président, Mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Guy Bénard Roche pour ne pas être trop long et pour les mêmes raisons que le rapporteur vous rassurer sur le fait que le fond Vert recouvre évidemment tout ce qui est Travaux de nature à isoler thermiquement les bâtiments et particulièrement les écoles bien sûr donc la position du gouvernement est défavorable. Merci madame la ministre, monsieur de la roche.

on l'a dit tout à l'heure dans la discussion générale qu'en fait, c'est quelque chose qui devient très compliqué et que par ailleurs, pour vous donner un an idée le faut le les décide, vous en parliez, mais la part de la dotation de la de la déciles alloués par l'État aux communes et dédié à la rénovation énergétique des bâtiments est estimé à moins de 10 % du montant total des déciles aujourd'hui donc, en fait, là, c'est le fait de cibler et de facilité était l'objectif de l'amendement. Et maintenu dans je mais on voit le 458 avec 2 avis défavorable qui est pour, qui est contre qui s'abstient, il n'est pas adopté le 642 monsieur Joly. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, cet amendement vise à mettre en place un fonds de maintien et de création des distributeurs automatiques de billets dans les communes rurales pour répondre aux difficultés d'accès aux services bancaires sur ces territoires, pour rappel des enjeux en 2019 rapport de la Banque de France, montrer que la quasi-totalité des communes de moins de 1000 habitants de était pas équipé en distributeurs de billets récemment le en juillet dernier, un état des lieux, là aussi, présenté par la Banque de France de, de, de démontrer la poursuite de la baisse du nombre de distributeurs de billets : moins 1000 distributeurs en une année ça participe à la désertification des territoires à travers cette désertification bancaire et en particulier dans les plus petites communes, la contrepartie, c'est la nécessité effectivement de faire ce 15 à 20 minutes de trajet pour accéder à ces services à un coût bien évidemment au regard de la flambée énergétique aujourd'hui, on mesure ce à quoi ça correspond, puis les contraintes environnementales aujourd'hui qu'on doit nécessairement prendre en compte les conséquences sont lourdes pour les populations de nos territoires moi digitalisée qui s'expose à un risque d'isolement et à une réduction de l'accès aux services bancaires sont pourtant essentiels dans la vie quotidienne, en particulier sur les territoires, or Hiro parle seulement, bien sûr, mais en particulier sur ces territoires d'où l'idée de créer ce fonds doté de 10 millions d'euros pour le maintien et la création des distributeurs de billets, merci. Si monsieur le rapporteur.

mais je me demande si on nous demandons s'il s'agit vraiment d'un service public qui doit être financé par des fonds publics et à l'heure actuelle 99 % de la population métropolitaine et est satisfaite, en étant à moins de 15 minutes il reste effectivement le 1 % qui qui pose toujours problème mais est-ce que un tel font ne créerait pas un un appel d'air en fait au au profit du monde bancaire, je crois qu'il vaut mieux qu'on qu'on continue à discuter avec lui pour, pour essayer de créer un réseau, voilà pourquoi je nous vous demandons à retrait sinon nous serions contraints défavorable. Si Madame la Ministre, de ma vie.

Il est pas plus si au surplus un jour on y ajoute les conséquences que ça dans la vie économique locale avec les petites transactions qu'il peut y avoir sont indispensables, on ne les change pas à travers des cartes bancaires, parce qu'il n'y a pas de de terminaux chez les agriculteurs chez des forestiers et il y a un service qui est véritablement offert grâce à cette possibilité de, de, d'échanger en espèces et il y a derrière un enjeu économique majeur sur des territoires dont la population aujourd'hui fait l'objet d'une paupérisation que l'on constate régulièrement merci. Si Monsieur le Président, mais c'est un vrai sujet pendant les 2 années qui se sont écoulées, nous avons vu que, avec les confinements successifs et tout ce qui s'est passé

je ne sais pas quelle sera l'issue du vote, mais il faudrait quand même que des mesures soient prises parce que, qu'il s'agit là de maths qui institutionnel également pour les personnes qui sont les miens ont les moins bien dotés, dans la mesure où il y a des personnes qui peuvent faire des virements, mais il y a beaucoup de personnes aussi qui sont victimes de l'illectronisme et qui ne peut pas faire systématiquement de et avoir de l'argent en espèce à certains moments, hé bien, c'est important pour les personnes qui n'ont pas d'autres possibilités. Oui, un mot pour dire que je j'approuve cette démarche pour les distributeurs automatiques, là, le milieu rural, on se retrouve un peu la dans la même problématique qu'évoquait il y a quelques jours, avec l'accès au haut les opérateurs là les banquiers à l'occurrence Estelle le distributeur automatique là où ça gagne beaucoup d'argent et refuse d'en mettre dans les communes rurales où il serait déficitaire, l'idée est bonne de financées par les crédits publics le les distributeurs automatiques le rural, moi pour ma part, je préférerai qu'il faut financer par les établissements bancaires à leur imposant pour tout distributeur à une zone urbaine, un distributeur jaune rural, il faut qu'ils prennent leur part. Ce Marc. de mon collègue de mon collègue Billac parce que, au-delà de l'investissement, c'est le fonctionnement annuel qui nous coûte, on a parlé avec les collègues, pour certains, 15000 euros par an, donc il faut plutôt passer par le fait d'imposer effectivement banques que dans un vaste plan où nous définir à quelle distance se trouvent les gens quelle distance temporelle, de façon à ce que nous puissions avoir un maillage complet du territoire a peut-être être passer par un autre système. Merci,

qui a les conséquences qui viennent d'être évoquées sur nos concitoyens, je partage aussi ce qu'a dit le rapporteur sur le fait que ça pourrait créer en le finançant par de l'argent public un appel d'air et que du coup les banques auraient tout d'un coup un intérêt à en installer davantage que ce qu'elles font, aujourd'hui, je crois qu'on touche là un point précis, c'est qu'on a besoin d'un réseau de service public, y compris bancaires qui pourrait, qui a été par le passé, assuré par la Poste et dont on voit qu'il nous manque aujourd'hui, et donc moi je suis assez partagé, j'aimerais pouvoir voter cet amendement qui répond à un besoin, mais en même temps il y répond, je crois, hein, parfaitement parce que ce qu'on ce qu'on a besoin, c'est un réseau de service public bancaire qui assumerait notamment cette mission-là. Si donc je le laisse voit cet amendement 642 avec 2 avis défavorable qui est pour.

Merci président, oui, ça peut paraître bizarre d'avoir un un amendement qui a trait aux CRS MNS, maître nageur sauveteur ici, mais en fait, oui, la formation et la rémunération des CRS n'est n'est pas rattachée au budget de cette mission les communes ont à leur charge de rembourser les frais de mission et de déplacements occasionnés par la participation des maîtres nageurs sauveteurs CRS à la sécurisation des plages des littoraux français cet amendement vise donc à accroître les crédits affectés à la dotation générale de décentralisation des communes afin de pérenniser ce dispositif alors pérenniser ce dispositif il y a lieu de d'être vraiment inquiet et cette un dispositif qui fonctionne, mais que le ministère de l'Intérieur grignote, année après année, nous avons de moins en moins de CRS MNS mis à disposition sur nos plages, alors oui, peut être, peut-on faire assurer par des jeunes, cette mission de sécurité dans la mer, il n'en reste pas moins que moi, j'ai vu beaucoup d'interventions dans l'Atlantique, nous avons un phénomène de de baïnes, qui fait que, il y a 2 ans, cette personne après une heure de lutte acharnée, ont pu être sauvés, ce n'était pas à la portée de tout le monde, et heureusement que ce sont les CRS MNS qui était à la manoeuvre, parce que je pense que nous aurions eu à déplorer beaucoup de victimes, parce que cela demande un entraînement intensif, simplement ils n'ont pas que cette mission en fait dans la mer, ils ont aussi la surveillance des plages parce que nous voyons de plus en plus de difficultés sur ces plages de sécurisation avec des bandes qui arrive et qui mettent à mal les touristes au ou les usagers des plages, alors que les CRS ont la possibilité, cette dissuasion avec l'arme

monsieur le président, madame la présidente, Delattre, évidemment vous avez exposé dès le départ que, a priori, vous n'étiez pas tout à fait dans la bonne mission en même temps, en essayant d'indiquer que les frais de déplacement, c'était peut être pas à la mission de sécurité, en tout cas ce n'est certainement pas la mission RCT, donc je vous demanderai le retrait qu'le soit bien clair sur le sujet je me dis quand même, on est dans un système où le ministère de l'Intérieur, si je comprends bien, prend en charge les CRS dans ces communes-là et ne prend pas en charge les frais déplacements mais, de mémoire, comme ça, on parle bien de communes littorales, on parle bien de communes con quand même quelques ressources, je me demande, je me demande vraiment si faut demander toujours à l'État plus vous voyez bon je pense que les communes littorales survivrait à prendre en charge ces frais déplacement en tout cas moi je suis prêt à devenir une commune littorale avec leur budget et de montagne ne t'inquiète pas, c'est la même chose pour les montagnes souvent et prendre de quelques frais déplacement à ce titre donc retrait bien sûr chers collègue. Si Madame la Ministre, même avis. Pour les mêmes raisons que monsieur le rapporteur, je demande à madame la sénatrice de l'air de bien vouloir retirer si dans le vote du Gouvernement sera défavorable, merci. Si. Madame la présidente,

parce que c'est important, on aura peut être un problème pour surveiller nos plages en 2024 puisqu'il a un retrait de de personnel pour mettre plus sur la capitale. Merci donc je mets aux voix l'amendement 399 avec 2 avis défavorable qui est pour.

les contraintes liées au fonctionnement de la DPV alourdissent la gestion de ces crédits, la répartition par enveloppes départementales tente à creuser les inégalités entre territoires selon les préfectures chargées de répartir les enveloppes de plus les communes éligibles à la DPV aurait été élargi sans que le montant de la dotation ne soient renforcées, cela a pour effet de mettre en difficulté les communes les plus précaires pour 2023, le budget est resté ça stables en autorisations d'engagement et a légèrement diminué en crédits de paiement 130 millions au lieu de 133, il est donc crucial pour lutter contre l'aggravation, la disparité des territoires de renforcer leurs moyens et le budget le le l'amendement propose un transfert de 500000 euros en fait. Et monsieur le rapporteur. c'est une demande de retrait puisque vous avez raison sur un point indiscutable, c'est que la dotation a été maintenu à 150 millions d'euros depuis 2017, ça c'est une évidence, cependant l'exécution en crédits de paiement, elle est toujours au crédit ouvert, disponible, donc pour l'instant il n'y a pas besoin d'argent supplémentaires sauf à montrer qu'il y a un besoin à ce moment-là je il y aurait sans doute un intérêt à augmenter à augmenter le montant donc demande de retrait. Merci madame la ministre. Juste pour compléter, monsieur le sénateur, les propos du rapporteur, simplement, il nous semble beaucoup plus raisonnables de traiter ce sujet en gestion au regard des faibles montants en jeu et je vous demande, nous aussi, au nom du gouvernement de retirer votre amendement. Merci monsieur B. Roche il est maintenu. Oui, les maths, je voulais juste préciser que le nombre de communes le périmètre à a augmenté par contre. Merci donc je mets aux voix le 463 et 2 avis défavorables qui est pour, qui est contre qui s'abstient, il n'est pas adopté, je me mettre aux voix le crée les les crédits de la mission Relations avec les collectivités territoriales figurant à l'état B je vous rappelle que la commission des finances, est favorable à l'adoption des crédits de cette mission, donc qui est pour. Qui est contre qui s'abstient ils sont adoptés, madame la ministre, est ce que j'ai oublié de vous demander le la levée du gage tout à l'heure pour les amendements 98 et 402 402 vous aviez émis un avis de sagesse sur celui de Monsieur Delcros et celui de la présidente de qui ensuite avait été Favre identique, vous êtes d'accord pour lever le gage. Pas de lever le gage, monsieur le président. Vous savez, gage d'accord, donc voilà. Je vais suspendre la séance, elle sera reprise à 14 heures 35 pour la suite de l'examen de la mission Relations avec les collectivités territoriales, la séance est suspendue.